Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues,

84 sont inscrites au réseau d'alerte des finances locales, 26 font l'objet d'un plan de redressement, 24 ont vu leur budget arrêté par le préfet en 2018 et 20 d'entre elles cumulent l'ensemble de ces critères d'alerte.

ce que votre gouvernement a su faire, monsieur le Premier ministre. En effet, celui-ci a diligenté rapidement, dès avril 2019, une mission confiée au député Jean-René Cazeneuve et à moi-même. Nous vous avons remis un rapport comportant 46 recommandations.

La dynamique d'ajustement des recettes a été vite enclenchée. C'est une très bonne chose car, dès cet exercice budgétaire, les communes des 5 DROM verront s'accroître le niveau de leur dotation de péréquation. Reste maintenant, pour parvenir à un véritable assainissement financier, à traduire dans les faits toutes les autres recommandations du rapport, notamment celles qui visent à améliorer la gestion des communes et à leur assurer un meilleur accompagnement. Je pense tout particulièrement à ces communes dont la situation rend parfois improbable, sinon impossible, un redressement financier sans soutien extérieur. Et il en existe quelques-unes ! Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple et peut-être un peu brutale, mais elle est à la hauteur des enjeux

Jacqueline Gourault, puisque c'est vous qui me répondrez, le 28 janvier dernier, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers professionnels annonçait mettre un terme à son mouvement social commencé il y a plus de sept mois. Cette annonce faisait notamment suite à votre décision d'engager un processus permettant une revalorisation de l'indemnité de feu, en portant son taux maximal de 19 % à 25 % d'ici à l'été prochain.

Le dynamisme de l'actuelle fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) allouée aux conseils départementaux dans le cadre du financement des SDIS ne saurait suffire. De nouvelles pistes de financement doivent donc être mises à l'étude. Une augmentation de la fraction de la TSCA allouée à nos départements en est Une modulation de la surcotisation, qui est versée par les employeurs et les pompiers, et qui est perçue par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour l'intégration de l'indemnité de feu dans le calcul des pensions, en est une autre. Madame la ministre, la prime de feu des pompiers n'avait fait l'objet d'aucune revalorisation depuis 1990. Sa réévaluation apparaît donc comme légitime et l'État doit accompagner les employeurs pour concrétiser cette ambition. Dans les Bouches-du-Rhône, où le directeur du SDIS est par ailleurs le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, nous savons, comme dans tous les départements français, combien la préservation de notre modèle de sécurité civile est essentielle. Nouvelles ressources, suppression des charges existantes, madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont vos pistes de travail pour dégager, à court terme, de nouvelles marges de manoeuvre auprès des SDIS et des collectivités concernées ?

des élèves séquestrés et cadenassés, d'autres passés à tabac, d'autres encore sanctionnés d'un zéro ou interdits de passer des épreuves, voire poursuivis en justice, des épreuves surveillées par des policiers : le baccalauréat version « nouveau monde » donne lieu à des scènes surréalistes Face au malaise grandissant, les seules réponses que vous apportez résident dans le mutisme et la répression. Pourtant, ce naufrage aurait pu être évité si vous aviez écouté les réserves émises, ici même, au Sénat, sur l'organisation des épreuves du contrôle continu

Par ailleurs, chacun sait ici que l'avenir de nos jeunes et de nos enfants est ce que nos concitoyens ont de plus précieux. Il faut entendre cette demande

principale innovation de la réforme du baccalauréat. Ces épreuves, qui compteront pour 30 % de la note finale du baccalauréat, se déroulent actuellement en classe de première. Cette version hybride entre contrôle continu et examen terminal est dénoncée tant par les enseignants que par les chefs d'établissement, les lycéens et leurs parents.

D'ailleurs, selon les membres du comité de suivi du nouveau bac, les E3C seraient « contraires à l'esprit de simplification de la réforme du bac » et des ajustements doivent être proposés. À plusieurs reprises, monsieur le ministre, nous vous avons alerté ici sur les difficultés qu'engendrerait toute précipitation dans l'application de votre réforme.

De jour en jour, les tensions s'accroissent et de nombreux établissements ont dû reporter les épreuves. Monsieur le ministre, il ne s'agit plus de minimiser les difficultés. Qu'attendez-vous pour reconnaître la réalité et corriger les errements de cette réforme ? La parole

Aujourd'hui, la pension moyenne des agriculteurs réunionnais est de 375 euros. Un quart d'entre eux perçoit moins de 100 euros. À ce bilan dramatique s'ajoute une inégalité criante avec la France

En 2018, alors qu'une proposition loi visant à revaloriser les retraites agricoles avait été adoptée par l'Assemblée nationale, son examen au Sénat avait été subitement bloqué par le Gouvernement au motif que ce sujet serait pleinement intégré à la réforme des retraites. Malheureusement, cet engagement de l'État semble aujourd'hui remis en cause et suscite naturellement de vives inquiétudes auprès des agriculteurs réunionnais et des représentations syndicales. La retraite universelle, oui ; mais pour les paysans d'outre-mer, non ! Monsieur le ministre, le Gouvernement compte-t-il respecter ses engagements en réparant cette inégalité entre La Réunion et la métropole ? La revalorisation des retraites agricoles fait-elle partie des priorités ? Le projet de loi que nous examinerons prochainement apporte-t-il des réponses

Il y a tout d'abord eu le rejet par Mme Pénicaud et les députés LREM de la proposition de loi portant à douze jours le congé pour décès d'un enfant. Quel manque spontané d'humanité Il y a eu le très sévère et, pour tout dire, inédit avis du Conseil d'État sur les retraites, qui a pointé du doigt les risques juridiques, l'absence de visibilité d'ensemble de la réforme, ainsi que le flou qui entoure son financement. Que d'inquiétudes

Le Président de la République a lui-même contribué à ce sentiment de flottement. Il s'est laissé immortaliser tout sourire avec un tee-shirt dénonçant les policiers, qui se sont sentis humiliés par celui qui devrait les protéger. outre, comment imaginer régler la difficile question de l'assimilation des jeunes générations issues de l'immigration, en rapprochant guerre d'Algérie et Shoah ? Monsieur le Premier ministre, vous qui conduisez le Gouvernement, nous attendons vos explications

mentionner un certain nombre d'autres indicateurs, dont je suis personnellement convaincu que vous vous satisfaites,

d'éléments qui ne gomment en rien ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur, mais qui doivent être mentionnés, car ils ne me semblent pas moins importants. les nombreux points que vous avez abordés, je voudrais rappeler un certain nombre de choses. Vous avez cité le cas de notre compatriote qui, après des propos critiques sur une religion, l'islam en l'occurrence, a été confrontée à des menaces de mort et, de ce fait, a dû faire l'objet d'une protection particulière et subir une déscolarisation forcée.

vont trouver un écho intéressant avec ceux qui ont été tenus par ailleurs. En vérité, monsieur le sénateur, le délit de blasphème n'existe pas ; la liberté de croire

savoir comment nous construisons la France, comment nous réparons des choses dont nous savons parfaitement, vous et moi, qu'elles fonctionnent mal depuis longtemps, comment, avec M. le ministre de l'éducation nationale, nous améliorons l'éducation

messieurs les sénateurs, que l'opération n'était pas simple à mener. Vous savez parfaitement que la France l'a conduite pour le compte de ses amis européens et que cette opération a été parfaitement réalisée. Cela fait, aussi, partie du tableau que vous auriez pu dresser, monsieur le sénateur, et, à mon sens, cela n'est pas moins important.

et que, « dans le contexte budgétaire actuel, une telle augmentation de charge n'est pas supportable ». Je vous remercie donc, madame la ministre, de bien vouloir m'expliquer comment cette mesure doit être financée.

et la caution que l'on donne à certaines caricatures. Lorsque l'on est Président de la République, investi des pouvoirs qui sont les siens, lorsque l'on est le garant des institutions et que, de ce fait, on dirige les forces de l'ordre et garantit l'ordre public, on ne se livre pas à des exercices de ce genre,

avec conviction, la défense des forces de police, qui sont sur le pont depuis l'affaire de, c'est-à-dire depuis cinq ans, et protègent notre démocratie de toutes les personnes, de plus en plus nombreuses dans le pays, qui menacent les valeurs de notre démocratie ?

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale. Les langues régionales constituent, pour la France, une richesse indéniable à bien des égards. La Délégation générale à la langue française et aux langues de France encourage leur préservation et contribue à leur valorisation. On comptait jusqu'à récemment plus de 92 000 élèves des premier et second degrés qui suivaient un enseignement en langues régionales, dont les trois quarts dans le service public d'éducation. Avec la réforme du baccalauréat, des classes de langues dites régionales ont fermé, tandis que d'autres sont en instance de fermeture ; des enseignants, démunis, se retrouvent avec moitié moins d'élèves que l'an passé. Dorénavant, une langue régionale prise en option facultative possède un coefficient minime, trois fois inférieur à celui des langues anciennes, ce qui représente 1 % environ de la note finale du bac. Il semble donc que la réforme du lycée soit un coup rude porté aux langues régionales. Pourtant, le président Emmanuel Macron déclarait, le 21 juin 2018 : « Les langues régionales jouent leur rôle dans l'enracinement qui fait la force des régions. Nous allons pérenniser leur enseignement. » Force est de constater que nous sommes aujourd'hui très loin de cet objectif On peut donc légitimement s'interroger sur la place qu'entend donner la France à ses langues minoritaires et régionales, pourtant qualifiées de richesse culturelle. En outre, est-il prévu de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et l'article 30 de la Convention internationale des droits de l'enfant protégeant le droit humain à pouvoir vivre dans sa langue ? La parole

Monsieur le ministre, je rappelle que, selon l'Unesco, 21 langues sont en danger ou sérieusement en danger en France, plus précisément aux Antilles, en Guyane et en Polynésie. et en Polynésie. Une langue est une part intrinsèque de l'être culturel. Il n'y a pas d'être sans culture. Donc porter atteinte à une langue régionale, c'est porter atteinte à l'existence même de l'être culturel. N'oublions pas que que la bête acculée n'accepte jamais d'être une victime expiatoire, mais livre toujours une farouche bataille pour survivre. Le message est clair ! La parole est à M. René Danesi, pour le groupe Les Républicains.

la difficulté d'accès aux soins devient une source d'inquiétude pour une partie grandissante de la population, surtout rurale et périurbaine. Dans certaines spécialités, il est courant d'attendre six mois pour avoir un rendez-vous. Certes, la médecine est quasiment gratuite, car prise en charge par la sécurité sociale et par les complémentaires santé. Mais la question de la santé dans les territoires se pose maintenant en termes d'équité. Il y a désormais une profonde injustice dans l'accès aux soins : cela est vrai pour la médecine de ville comme pour l'hôpital. Les pouvoirs publics, et vous n'avez pas fait exception à la règle, ont accumulé les plans contre les déserts médicaux. Mais ces plans sont sans efficacité, car ils ne traitent pas les causes du mal. On y retrouve des incitations financières, d'ailleurs souvent à la charge des communes, mais on y trouve surtout la bureaucratisation et la fonctionnarisation rampante de la médecine. À ceux qui s'alarmaient d'une situation devenue intenable, vous avez répondu par la suppression du, c'est-à-dire la suppression de la limitation du nombre des médecins formés. Cette suppression était présentée comme la solution au problème. Mais, dans les faits, les facultés de médecine, soucieuses de la qualité des formations, ont d'ores et déjà annoncé qu'elles n'avaient pas les moyens d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine. Madame la ministre, l'avenir de la médecine nécessite une vision stratégique. Les déserts médicaux ne sont que le symptôme du déclin de notre médecine de santé. Mes questions sont donc très simples. Êtes-vous prête à abandonner les fausses solutions qui n'ont cessé de dégrader la situation ? Êtes-vous prête à réformer vraiment, en repensant l'actuelle gouvernance asphyxiante de la santé en France, en démontrant votre confiance dans l'exercice libéral de la médecine par sa revalorisation ?

visent à apporter des solutions. La fin du ne représente qu'une petite partie de ces solutions. Elle a pour objet principal, non pas tant d'accroître le nombre d'étudiants en médecine, même s'il est possible de le faire un peu, mais surtout de diversifier le profil des étudiants et des territoires dont ils sont issus.

Tout leur est offert pour répondre à leurs besoins d'un exercice pluriprofessionnel, car la solution viendra de la délégation d'un certain nombre de tâches à d'autres professionnels, qui peuvent être extrêmement compétents,

Ma question s'adressait à M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Je tiens à y associer pleinement ma collègue Valérie Létard, sénatrice du Nord. Le 6 février dernier, la Commission européenne rejetait la fusion entre Alstom et son concurrent allemand, Siemens. et des finances avait alors qualifiée d'erreur économique et de faute politique, était justifiée par la commissaire européenne à la concurrence en raison de la réduction de la pression concurrentielle qu'une telle fusion aurait entraînée. Un an après, le groupe français envisage désormais l'acquisition des activités ferroviaires du canadien Bombardier, actuellement en grande difficulté financière. Une telle acquisition aurait de nombreux intérêts pour notre groupe tricolore, en ce qu'elle en ferait véritablement un champion du ferroviaire, pesant près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, présent sur de nombreux marchés étrangers et pour des gammes de produits complètes. M. le ministre défend un assouplissement des règles européennes afin d'introduire la prise en compte des intérêts stratégiques européens, et alors qu'en décembre dernier la nouvelle Commission européenne a annoncé sa volonté de réviser les règles de la concurrence européenne, envisage-t-il qu'une telle opération stratégique puisse, elle aussi, subir un veto de la Commission européenne, au nom de la concurrence ? Comment compte-t-il défendre les intérêts industriels de notre pays et de cette entreprise à Bruxelles ? Enfin, quelles garanties en termes d'emploi peut-il apporter pour nos territoires, afin que les emplois industriels ne constituent pas une variable d'ajustement d'un tel rapprochement, par ailleurs

Nous avons eu, et c'est de notoriété publique, une divergence avec la Commission européenne dans l'évaluation de la criticité et de la faisabilité de la fusion entre Alstom et Siemens.

d'État auprès de la ministre des armées, nos armées sont engagées dans des opérations qui s'inscrivent dans la durée. Elles doivent disposer de la meilleure technologie. souhaite promouvoir prioritairement les technologies françaises et les coopérations européennes. C'est une bonne chose ! La France compte, dans le domaine de la défense, de grands groupes, mais aussi des PME, voire des start-up, souvent plus vulnérables. La compétition fait rage entre les grandes puissances. Nous devons donc conserver nos compétences pour l'avenir de nos industries et celui de nos opérations. Pourtant, nous constatons avec inquiétude l'intérêt que suscitent à l'étranger, notamment aux États-Unis, quelques entreprises françaises de technologies sensibles. Ces précieuses pépites attirent souvent les convoitises. Certaines sont déjà passées sous pavillon étranger ; d'autres seraient en passe de l'être. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre souveraineté

Aujourd'hui, le temps s'est écoulé, et j'entends qu'aucune solution industrielle française ne semble se dégager, quand des acheteurs non européens semblent déjà prêts. Il y a donc urgence à agir.

le plan de l'autonomie stratégique européenne. Le budget de la défense européen, le Fonds européen de la défense, sera là aussi un atout majeur. Entre 2021 et 2027, 13 milliards d'euros seront ainsi dévolus à la recherche, à l'innovation,

Samedi dernier, le quotidien a fait paraître sa dernière édition, après cinquante-six ans d'existence. Le tribunal de commerce de Fort-de-France a en effet prononcé la liquidation judiciaire du journal sans poursuite d'activité. Je pense tout d'abord naturellement aux 235 salariés et aux familles impactées : 112 salariés en Martinique, 99 en Guadeloupe et 24 en Guyane, qui travaillaient dans les rédactions et s'inquiètent légitimement pour leur avenir. Toutes proportions gardées, à l'échelle nationale, c'est l'équivalent d'un millier de personnes licenciées dans la plus grande indifférence. Fondé en 1964, était diffusé à environ 35 000 exemplaires en Martinique, 25 000 en Guadeloupe et possédait une déclinaison pour la Guyane sous le titre. Le journal Le journal servait également de lien avec leur territoire pour tous les Guadeloupéens et Martiniquais vivant à Saint-Martin. La disparition du journal laisse donc ces trois territoires sans quotidien d'envergure, alors que le Président de la République, à l'occasion de ses voeux à la presse le 16 janvier dernier, s'était engagé à soutenir la presse d'outre-mer en difficulté. Monsieur le secrétaire d'État, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Premièrement, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi l'aide à la presse hexagonale ne s'applique pas à la presse ultramarine ? Deuxièmement, ne pensez-vous pas qu'au regard des situations de plus en plus dégradées dans nos territoires les tribunaux devraient s'attarder plus longuement sur les sur les possibilités de reprise ? a été liquidé en dix minutes chrono ! Enfin, puisqu'il semblerait que ces difficultés iront en s'amplifiant au regard de l'essor du numérique, comment comptez-vous garantir un avenir pour la presse écrite ? La parole

prononcé la liquidation. Il faut mesurer, comme vous l'avez dit, l'ampleur de cette décision, d'abord pour les 235 salariés concernés. Cette annonce intervient alors que l'ensemble des ministères s'était mobilisé depuis plusieurs mois pour accompagner l'éditeur dans la recherche d'une solution permettant le maintien des trois publications.

leur reconversion professionnelle, de la création de nouvelles activités liées à la filière média ou de diversification. Plus globalement, le ministère de la culture mobilisera ses dispositifs en fonction du type de projet présenté pour permettre l'émergence de nouveaux médias dans les Antilles. Les différentes aides à la presse, qu'il s'agisse d'aides au fonctionnement ou à l'investissement, générées par le ministère de la culture, sont ouvertes à l'ensemble des titres de presse. Il apparaît que, compte tenu du modèle d'affaires un peu particulier des types de presses dans les outre-mer, ceux-ci bénéficient un peu moins des aides à la presse que sur le territoire national. Je veux ici vous annoncer que le ministère de la culture va dans les prochains mois modifier les conditions d'attribution de plusieurs aides pour les titres ultramarins, afin de rétablir une forme d'équité de traitement. Les services du ministère de la culture accompagneront étroitement tous les projets de presse qui naîtront sur ces territoires, afin d'y restaurer un vrai pluralisme de l'information.

Jasmin, pour le groupe socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale. Monsieur le ministre, je souhaite relayer ici les craintes des parents d'élèves et des enseignants de la Guadeloupe sur l'avenir de l'enseignement public. L'ensemble du système scolaire et universitaire y est désormais en danger, et les dernières annonces de votre gouvernement concernant la suppression de postes dans de nombreuses académies ont suscité ont suscité l'émoi des parents d'élèves et des enseignants. Par ailleurs, les déclarations inquiétantes d'un ancien ministre concernant la mutation secrète d'enseignants supposés pédophiles en outre-mer suscitent également l'émoi, la consternation et des interrogations au sein de la population. Au moment où je vous parle, et ce depuis plusieurs semaines, 90 % des écoles et des établissements scolaires de l'archipel sont bloqués par un mouvement de grève. Au-delà de la consternation des enseignants à votre réforme des retraites, les revendications en Guadeloupe portent sur les moyens accordés par l'État dans le cadre des politiques éducatives mises en place sur le territoire. Les conditions d'enseignement se dégradent considérablement. La qualité de l'apprentissage, ainsi que l'accompagnement des enfants en situation de handicap sont au coeur du mécontentement, amplifié par l'annonce récente de la suppression de 72 postes d'enseignants à la rentrée prochaine, après 86 suppressions en 2019 et Une rencontre entre le recteur et les grévistes a eu lieu vendredi dernier, date d'un début de dialogue et de la présentation d'un moratoire. l'inquiétude demeure face à la dégradation des conditions d'exercice et à la réduction drastique incompréhensible des moyens, notamment pour la prise en charge d'enfants en difficulté. Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous pour les enfants en situation de handicap, et plus particulièrement pour répondre au moratoire sur les cinq ans à venir afin de garantir la qualité de l'enseignement et rassurer les parents d'élèves, la population et avant tout les enseignants ? La parole La parole est à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le de l'éducation en Guadeloupe. Je m'en réjouis parce que nous avons évidemment beaucoup de choses à nous dire sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. Vous me posez plusieurs questions, auxquelles je vais essayer de répondre en deux minutes.

sera amélioré, comme c'était déjà le cas lors de la rentrée précédente. Aujourd'hui, le taux d'encadrement en éducation prioritaire en Guadeloupe est de 17,6, pour plus plus de 20 à l'échelle nationale ; rappelons aussi que 65 % des écoles en Guadeloupe ont moins de 22 élèves par classe. Le taux

Monsieur le ministre de l'éducation nationale, ma question porte elle aussi sur les épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat, qui ont commencé le 20 janvier et se dérouleront jusqu'à fin février. Ces dernières, cela a été rappelé, suscitent des manifestations et des blocages organisés par des élèves, des professeurs et des syndicats. Dimanche 2 février, 166 annulations et reports d'épreuves avaient été signalés, 51 épreuves où tous les élèves n'ont pas pu composer et 148 lycées où les épreuves ont été sérieusement perturbées. Mon département, la Haute-Savoie, n'est pas épargné : des épreuves ont été annulées, notamment aux lycées Berthollet et Fauré à Annecy, et au lycée Lachenal à Argonnais, tandis que d'autres lycées ont vu leurs épreuves perturbées par les manifestations, comme le lycée des Glières à Annemasse, le lycée Baudelaire à Annecy et le lycée Charles-Poncet à Cluses. Nous sommes donc en présence d'épreuves annulées ou reportées,

Les élèves et leurs parents ne savent pas quelles seront les modalités pour les examens annulés, ni si le barème sera adapté pour les épreuves ayant été perturbées, ou si ces dernières seront repassées ultérieurement. Des élèves n'ayant pas pu passer leurs épreuves risquent un zéro et les rattrapages, alors qu'ils ont simplement eu la malchance de ne pas réussir à entrer dans leur établissement avant le début des blocages. J'ai reçu de nombreuses vidéos en attestant. Cette situation est anxiogène pour les élèves et leurs parents, qui ne connaissent pas les solutions qui seront mises en place pour pallier ces perturbations. De nombreux témoignages font état d'une dégradation de la santé mentale des élèves, qui sont dans l'incompréhension totale et extrêmement angoissés par rapport à ces épreuves. Sachant que ces questions sont largement laissées à l'appréciation des chefs d'établissement, cela ne fait qu'ajouter à l'incertitude des élèves. Je vous demande donc, monsieur le ministre, si vous comptez donner des consignes spécifiques aux chefs d'établissement afin d'homogénéiser au mieux ces épreuves au niveau national. Je vous demande également si des mesures spéciales seront mises seront mises en place afin que les épreuves n'ayant pas encore eu lieu puissent se dérouler le plus sereinement possible. La

extérieurs, qui ne doivent pas commettre des actions illégales. S'agissant des élèves, notre attitude est évidemment dictée par la plus grande bienveillance. Nous allons regarder, établissement par établissement, comment éviter

pour. Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle, en application de l'article 16 , alinéa 2, du règlement, la proposition de création d'une commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'accélération et de simplification de

Conformément à la décision de la conférence des présidents, la désignation des trente-sept membres de cette commission spéciale aura lieu en séance publique, demain, à L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols. En application de l'article 8 , alinéa 5, du règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par le règlement. L'ordre du jour appelle, à la demande du groupe La République En Marche, l'examen de la proposition de résolution relative aux enfants franco-japonais privés de tout lien avec leur parent français à la suite d'un enlèvement parental présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par M. Richard Yung et plusieurs de ses collègues (proposition n° 29). Dans la discussion générale, la parole est à M. Richard Yung,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a tout juste neuf ans, la Haute Assemblée adoptait à l'unanimité une proposition de résolution appelant les autorités japonaises à garantir le respect du droit des enfants franco-japonais séparés de l'un de leurs parents. Nous avions lancé cet appel après avoir constaté que des enfants binationaux étaient privés de tout contact avec leur parent français à la suite d'un enlèvement commis par leur parent japonais. Le constat dressé en 2011 est malheureusement toujours d'actualité. Voilà quelques jours, deux enfants franco-japonais ont été enlevés par leur mère japonaise. Ils ont subi le même sort que les enfants d'un ressortissant australien qui a récemment passé quarante-cinq jours en garde à vue avant d'être condamné à six mois de prison avec sursis. Son tort ? Avoir tenté de voir ses enfants après le passage d'un violent typhon. La sévérité de la peine infligée à ce père a conduit les autorités australiennes à exprimer leur préoccupation quant à l'application, par les juges japonais, du principe non écrit dit « de continuité », qui consiste à attribuer systématiquement l'autorité parentale et la garde exclusive de l'enfant au parent ravisseur. Au Japon, le partage de l'autorité parentale et la garde alternée n'existent pas. De plus, l'exercice du droit de visite dépend du bon vouloir du parent qui a la garde de l'enfant. Il suffit en effet à ce dernier de dire à son ex-conjoint que l'enfant est malade ou ne veut pas le voir pour annuler une visite. Il suffit effectivement de faire pression sur l'enfant. On m'a raconté le cas d'un enfant qui certes

Le parent ravisseur profite de l'absence de l'autre parent pour vider le logement. Il se réfugie ensuite chez ses parents avant d'accuser son conjoint de violences conjugales. Au Japon, une simple déclaration suffit et aucune enquête n'est menée.

Lorsque le couple est établi à l'étranger, l'enlèvement a généralement lieu lors du séjour temporaire au Japon de l'un des parents. À cet égard, je condamne fermement les propos qui ont été tenus par un groupe d'avocats japonais à l'occasion d'un séminaire organisé à Paris le 15 mai 2018. Ces avocats avaient alors expliqué à des Japonais résidant en France comment « légaliser » l'enlèvement d'un enfant depuis notre territoire. Nous ne savons pas précisément combien d'enfants japonais se trouvent actuellement privés de tout contact avec l'un de leurs parents.

Les plus nombreux sont des enfants américano-japonais. Pour ce qui est des enfants franco-japonais, onze dossiers sont actuellement suivis par le Quai d'Orsay. Ce nombre relativement faible ne reflète cependant pas la réalité. de nombreux cas n'ont pas été portés à la connaissance des autorités diplomatiques et consulaires, soit parce que le parent concerné ignore qu'il peut s'adresser au consulat,

En 2014, le Japon a adhéré à la convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. L'entrée en vigueur de cette convention n'a malheureusement pas permis de résoudre certaines situations douloureuses, qui persistent par des pratiques installées dans les moeurs, mais aussi par l'application de la législation japonaise en matière de droit de la famille. Des décisions judiciaires prises en vertu de la convention de La Haye ne sont pas exécutées ou le sont difficilement. Aussi surprenant que cela puisse paraître,

Autrement dit, le juge s'est prononcé et il ne se passe rien ! Les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne représentés au Japon ont, dans une démarche commune, signalé à plusieurs reprises au gouvernement nippon « l'importance de l'exécution des décisions des tribunaux japonais ». Au regard de ce constat, il apparaît nécessaire d'encourager les autorités japonaises à prendre des mesures urgentes pour garantir le respect des droits fondamentaux des enfants, notamment franco-japonais, au centre d'un conflit parental. Le Président de la République s'est engagé à agir en faveur des parents qui vivent ces situations de détresse et en a parlé au Premier ministre lors de sa visite officielle au Japon au mois de juin dernier. J'espère qu'il sera répondu favorablement à sa demande de rétablir en particulier le comité consultatif franco-japonais relatif à l'enfant au centre d'un conflit parental,

D'autres chefs d'État ont interpellé les autorités japonaises. Des mesures préventives ont été prises récemment par l'Allemagne et l'Italie.

que la Haute Assemblée a récemment adopté une résolution européenne et un avis politique visant à faire en sorte que l'Union européenne s'exprime avec force et d'une seule voix. Je forme le voeu que le Parlement européen adopte rapidement, peut-être ce mois-ci, une proposition de résolution allant dans le même sens que celle que nous allons, je l'espère, adopter

et de la société japonaise en général. Nous sommes donc mus par des sentiments d'amitié et souhaitons voir le Japon évoluer dans le sens que nous indiquons. vise surtout à soutenir les efforts diplomatiques déployés par la France et ses partenaires européens. À cet égard, je tiens à remercier notre ambassadeur à Tokyo et son équipe de leur implication dans ce dossier particulièrement complexe et douloureux. Je tiens aussi à saluer le travail mené par les associations, notamment l'association Sauvons nos enfants Japon, qui apporte un indispensable soutien humain et juridique aux parents privés de tout contact avec leurs enfants. enfin de remercier mes soixante-dix-sept collègues cosignataires de cette proposition de résolution. Pour conclure, je souhaite vous informer que notre vote est très attendu par les associations japonaises de défense des parents en situation de divorce

Notre vote est également attendu par des parlementaires japonais, de la majorité comme de l'opposition, qui cherchent à faire évoluer la législation nippone. Plusieurs d'entre eux m'ont dit vouloir s'appuyer sur nos résolutions pour faire valoir leur point de vue auprès de leurs collègues et du gouvernement Abe, même si ce n'est pas si facile. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à

les paroles insoutenables de Stéphane Lambert, père français dont l'enfant a été enlevé par sa mère en 2015. Ce témoignage traduit l'importance du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Il traduit aussi la situation de nombreuses Françaises et de nombreux Français faisant face à des situations d'enlèvement parental. Je souhaite remercier le groupe La République En Marche de nous permettre de nous exprimer sur le sujet, en particulier Richard Yung. Chacun, dans cet hémicycle, sait l'engagement et le dévouement dont il fait preuve depuis des années aux côtés des parents confrontés à cette situation. Je souhaite également saluer la commission des affaires européennes du Sénat ainsi que Véronique Guillotin pour leur travail conjoint. Un rapport et une proposition de résolution européenne traitant des enlèvements d'enfants euro-japonais par leur parent japonais ont dégagé des pistes de réflexion. Les institutions européennes ont d'ailleurs été saisies de ce sujet. La proposition d'une nouvelle rencontre entre ambassadeurs des États membres de l'Union européenne et les autorités japonaises, formulée dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui, est à mes yeux essentielle. Nous devons développer un dialogue constructif sur ce point. En effet, ce problème, qui n'est pas nouveau, ne constitue pas non plus une particularité française. De nombreux pays, à commencer par les États-Unis, y sont également confrontés. Des ressortissants italiens, australiens, ou encore britanniques font face à ce traumatisme. Ce fait concerne des dizaines de milliers d'enfants par an. La bataille juridique qu'imposent ces situations est très souvent vécue comme un parcours du combattant pour le parent souhaitant retrouver son enfant. De nombreuses actions ont été menées dans le monde : récemment, un cabinet français a porté ce sujet devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. La proposition de résolution que nous étudions aujourd'hui retrace les particularités du droit de la famille japonaise. Nous l'avons déjà souligné, la non-reconnaissance de l'autorité parentale partagée, d'une part, l'impossibilité d'un droit de garde alternée, d'autre part, en sont les deux points clés. Le principe de continuité, aussi mis en exergue, s'ajoute aux difficultés. À cela, la résolution oppose un champ lexical ne laissant aucun doute sur la nature du problème et les effets sur les enfants concernés, qui « se retrouvent privés d'une part essentielle de leur identité », souffrent d'un « déficit affectif susceptible de nuire à leur développement personnel

faire, et nous observons que les trois points que je viens d'évoquer- l'autorité parentale, la garde alternée et le principe de continuité -ne sont pas concernés par l'évolution de la loi. Or ils représentent une partie de la solution.

La première, découlant du nécessaire dialogue entre la France et le Japon, vise la création d'un poste de magistrat de liaison à l'ambassade de France au Japon. Cette liaison me semble primordiale, d'autant plus qu'un tel magistrat existe déjà auprès de l'ambassade du Japon en France. Ce serait un moyen supplémentaire de faciliter la gestion de divers cas entre nos deux pays. La deuxième suggestion est le rétablissement du comité consultatif franco-japonais relatif à l'enfant au centre d'un conflit parental. Ce comité n'est plus actif depuis 2014, mais il pourrait permettre un dialogue plus constructif et plus efficace. Enfin, le dernier point de cette proposition de résolution que je souhaite mettre en avant est la sensibilisation de nos magistrats. Les conflits de droit international privé sont très complexes, et nous devons prendre en compte tous leurs aspects. D'autres points de ce texte auraient pu être soulevés. Il est important que cette question soit abordée de manière régulière aux échelons européen et international. Je suis convaincu que la création d'une liste européenne des pays qui ne respectent pas leurs obligations relatives à la convention de La Haye serait une bonne chose. Les droits fondamentaux des enfants et des parents doivent être respectés et préservés. Le lien des enfants avec leurs parents est à bien des égards une nécessité et participe au bien-être La France et le Japon, dont les liens sont forts depuis de nombreuses années, doivent poursuivre leurs efforts de dialogue pour trouver des solutions aux problèmes des enlèvements parentaux.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, en préambule, j'associe à cette intervention M. Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger qui, durant plusieurs années, a porté ce combat avec détermination. Une affaire récente a particulièrement marqué l'opinion française. Ce fait divers est aujourd'hui connu de tous : initialement, il s'agit d'une histoire familiale, donc personnelle et intime, mais elle s'est soldée par un déchirement humain et un écho médiatique retentissant. mariage en 2008 à Toulouse, un couple décide de s'installer au Japon. En 2015, son fils, Louis Kudo-Verhoeven, naît à Tokyo. Deux ans plus tard, alors qu'elle est en France avec son fils, la mère souhaite divorcer et ne plus rentrer au Japon. Le 26 décembre dernier, le petit Louis, âgé de 4 ans, est reparti dans sa terre natale, après une demande de retour de son père. Le départ a eu lieu entouré de gendarmes et sous l'oeil des caméras. La mère de Louis- française -a pourtant apporté les preuves qu'elle n'aurait vraisemblablement plus la possibilité de voir son fils jusqu'à la majorité de celui-ci, fixée au Japon à 20 ans. En effet, elle ne possède pas de visa lui permettant de résider au Japon, la législation nippone étant extrêmement restrictive en termes d'obtention de ce type de document, notamment durant une procédure de divorce. l'autorité parentale partagée n'existant pas en droit japonais et l'autorité exclusive ayant été octroyée par la justice au père japonais, la mère de Louis ne pourra très probablement pas bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent, puisque ce statut est directement lié à l'autorité parentale. En un mot, la situation est inextricable. Louis risque donc de se voir coupé de tout lien avec sa mère et sa famille française, alors même qu'il était scolarisé en France et menait une vie tranquille et sans histoire, que tous les enfants de 4 ans devraient avoir. Louis n'est malheureusement pas le seul enfant dans ce cas, et les médias font régulièrement état de la situation de parents désespérés, en France, mais aussi chez nos voisins. Une telle séparation « légale » d'un parent et de son enfant constitue un véritable traumatisme pour toutes les personnes impliquées, en premier lieu pour les enfants eux-mêmes.

Je sais que son combat est ancien ; je veux l'assurer de tout le soutien du groupe socialiste dans sa démarche. En visite au Japon le 27 juin 2019, le Président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé à agir en faveur de ces pères français et, plus largement, des parents non japonais. Il a évoqué les « situations inacceptables » vécues par des enfants binationaux et leur parent français avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe. Nous saluons cette prise de position officielle, car le besoin concret de la France se fait sentir, afin que parents et enfants ne soient plus privés les uns des autres. les uns des autres. Le Japon est un pays ami, un allié, avec lequel ont été passés de très nombreux accords dans tous les domaines, des échanges commerciaux à la fiscalité en passant par la sécurité sociale. Dès lors, pourquoi est-il si difficile de s'entendre sur ce sujet si sensible pour les familles concernées ? Le plus absurde est que ces drames perdurent malgré la ratification par le Japon, le 24 janvier 2014, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, puis la création, à Tokyo, d'une autorité centrale chargée d'assister les parents d'enfants enlevés. En effet, c'est sur une adaptation en droit japonais de la convention de La Haye, favorable aux parents japonais, que se fondent les décisions des juridictions nippones. À cela s'ajoute l'incapacité de la justice à faire appliquer les rares ordonnances de retour qui ont été prononcées à ce jour. Il est impératif que les jugements français soient respectés par les juridictions japonaises, et que les divorces prononcés par les tribunaux français soient intégralement retranscrits là-bas. Le ministère des affaires étrangères a plusieurs fois indiqué qu'une réflexion spécifique aux conflits familiaux au Japon était menée en lien avec les autorités japonaises, afin d'explorer les possibilités de faciliter la résolution de ces situations douloureuses. Il s'agit d'obtenir des autorités japonaises la mise en place d'une instance de dialogue, fonctionnant sur le modèle de celle qui a été créée en 2009, puis supprimée après l'adhésion du Japon à la convention de La Haye en 2014. réflexion, madame la ministre ? Bien sûr, la France n'est pas le seul pays concerné par de telles situations. Au mois de janvier 2018, dans le cadre du rapport du groupe de travail des Nations unies sur l'examen périodique universel sur le Japon, le Canada et l'Italie ont questionné le Japon sur la mise en place de ces mécanismes juridiques le contraignant à faire respecter le droit de visite et permettant d'entretenir des liens réguliers avec les deux parents. Au mois d'avril suivant, les États-Unis ont inscrit le Japon dans la liste des pays qui ne respectent pas la convention de La Haye de 1980. Malgré ces actions symboliquement fortes, la situation ne s'améliore pas- ou si peu ! La mention d'une coopération européenne dans la proposition de résolution est donc la bienvenue. Il nous faut en effet peser de tout notre poids diplomatique pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Nous espérons vivement que le Gouvernement se saisira véritablement de la question, afin que cette initiative soit suivie d'effets.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je remercie tout d'abord M. Richard Yung d'avoir présenté une proposition de résolution relative aux difficultés rencontrées par les parents français d'enfants franco-japonais. Que se passe-t-il en cas de divorce ou de séparation de couples franco-japonais ? La réponse est simple : lorsque les enfants sont emmenés au Japon par le parent japonais, le parent français court le risque de ne plus jamais les revoir. En effet, selon les principes du code civil japonais, l'autorité parentale partagée n'est pas reconnue. Traditionnellement, le foyer est constitué des deux parents et du ou des enfants. Si le couple divorce, l'enfant n'« appartient » plus qu'à un des deux parents. Contrairement à la France, les tribunaux japonais refusent de reconnaître les jugements de divorce prononcés à l'étranger. Ils n'hésitent pas à réattribuer la garde et l'autorité parentale au parent japonais lorsqu'il a enlevé les enfants et les a ramenés au Japon, même si un tribunal français les avait précédemment placés sous la responsabilité de l'autre parent. Lorsque ces faits d'enlèvement se produisent à l'intérieur même du Japon, les juges protègent les parents japonais et entérinent les enlèvements. le droit de visite ne fait pas partie des moeurs du pays. Lorsqu'un parent français l'obtient, ce droit demeure très sévèrement encadré et soumis au bon vouloir du parent japonais. Par ailleurs, les autorités japonaises ne mettent pas en oeuvre les ordres de retour d'enfants binationaux dans un autre pays. Les agents chargés de la mise en exécution des ordonnances de retour refusent d'intervenir rapidement et par la force dans ces affaires civiles et familiales au motif qu'elles relèvent de la vie privée. Le 21 décembre, la Cour suprême du Japon a même annulé plusieurs ordonnances de retour préalablement rendues en faveur de James Cook, un Américain, père de quatre enfants enlevés par leur mère japonaise, ce qui donne un redoutable signal aux parents privés de leurs enfants. La loi japonaise ne punit pas l'enlèvement parental. Le Japon n'applique pas l'article 9-3 de la convention relative aux droits de l'enfant, dite convention de New York, qu'il a signée le 22 avril 1994- voilà quinze ans cet article dispose : « Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les parents français qui tentent de faire reconnaître leurs droits sont parfois arrêtés pour harcèlement, éventuellement soupçonnés de tentative d'enlèvement de l'enfant et placés en garde à vue pendant de nombreux jours. Certains ont été tellement désespérés de ne pouvoir entrer en contact avec leurs enfants qu'ils en sont venus au suicide. Le drame d'Arnaud Simon a ému la communauté franco-japonaise. L'ambassadeur Philippe Faure a publié le communiqué suivant M. Simon avait fait part récemment à la section consulaire de notre ambassade à Tokyo des difficultés qu'il éprouvait pour rencontrer son fils, et il est très probable que la séparation d'avec son enfant a été un des facteurs déterminants d'un geste aussi terrible. Ceci nous rappelle à tous, s'il en était besoin, la souffrance des 32 pères français et des 200 autres cas étrangers, recensés par les autorités consulaires comme étant privés de fait de leurs droits parentaux. le président Macron a rencontré les parents français dont les enfants franco-japonais ont été enlevés par leur parent japonais. Il a déclaré : « Il y a un droit japonais, qui est très différent du nôtre, mais il y a des situations de détresse qui sont absolument inacceptables. [Nous ferons] tout pour être aux côtés de [ces parents]. Il a précisé avoir évoqué ce problème avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser le résultat de ce soutien présidentiel ? Par-delà les formules diplomatiques, y a-t-il eu des résultats concrets ? Il est essentiel que nos consulats dispensent le maximum d'informations aux nouveaux résidents au Japon sur les spécificités de la loi japonaise en matière de divorce et d'autorité parentale. Je salue la mobilisation exceptionnelle de nos trois conseillers consulaires, Thierry Consigny, Evelyne lnuzuka et François Roussel, pour sensibiliser et accompagner nos compatriotes. Plusieurs associations, telles que Sauvons nos enfants Japon et SOS Parents Japan, effectuent un intense travail de sensibilisation politique et médiatique. Allez-vous, madame la ministre, soutenir l'action méritoire de ces associations ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution vise à résoudre une question difficile à plus d'un titre : difficile, car elle touche aux droits des enfants, en l'occurrence des enfants issus de couples franco-japonais qui, à la suite d'un divorce ou d'une séparation, se retrouvent privés de tout contact avec leur parent français difficile également, car elle relève de la souveraineté d'un État aux traditions juridiques et culturelles bien différentes de celles que nous connaissons dans nos sociétés occidentales. En effet, j'ai pu le mesurer lors de mes déplacements au Japon et au cours de mes échanges avec des parlementaires japonais, le gouffre culturel d'abord, judiciaire ensuite, qui nous sépare dans le traitement de ces affaires familiales est réel et profond. J'ai souvent été très surprise de constater que ces situations étaient tout à fait normales pour de nombreux Japonais, qui ne parvenaient pas à mesurer notre incompréhension devant ce qui représente pour nous une injustice flagrante. C'est un point que j'estime important : ces séparations douloureuses ne concernent pas seulement les couples binationaux ; elles sont au contraire profondément inscrites dans la société japonaise et touchent en premier lieu les familles japonaises, dont les séparations, lorsqu'elles ont lieu, sont, de notre point de vue, aussi violentes. Cette différence culturelle qui nous oblige à la prudence pour ne pas heurter la sensibilité de la partie japonaise, ne doit cependant pas nous empêcher de défendre avec force le droit de nos ressortissants. Je tiens à rendre hommage aux associations comme Sauvons nos enfants Japon, dont l'engagement continu auprès des parents français doit être salué. Le Sénat a toujours été sensible à cette question en 2011 déjà, nous avions adopté à l'unanimité une proposition de résolution destinée à appeler l'attention des autorités nippones sur la nécessité de reconnaître aux enfants franco-japonais au centre d'un conflit parental le droit de conserver des liens avec chacun de leurs parents. Notre diplomatie joue également un rôle important. Le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a multiplié les interventions, tout comme notre poste diplomatique au Japon, dont l'action auprès de nos ressortissants et de la partie japonaise est plus que précieuse. Néanmoins, il serait important qu'à l'avenir les visites consulaires soient rendues réellement effectives. En effet, actuellement, lorsqu'un enfant français est retenu au Japon, l'ambassade française peut uniquement solliciter une visite auprès du parent japonais, qui est libre de la refuser, ce qui, malheureusement, se produit dans la majorité des cas. D'autres États sont touchés et tentent, eux aussi, de sensibiliser le Japon à cette question. Je pense notamment aux États-Unis, dont la Chambre des représentants a adopté une résolution en 2010 et dont le département d'État a, en 2018, choisi de classer le Japon parmi les pays qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de La Haye. des Nations unies, par l'intermédiaire de son comité des droits de l'enfant, s'est également penchée sur les manquements du Japon à ses obligations conventionnelles et a fait récemment, le 1 février 2019, des recommandations aux autorités japonaises. Toutes ces démarches ne sont pas restées vaines, et le Japon a dernièrement pris des mesures qui, si elles ne sont pas spectaculaires, vont au moins dans le bon sens. Nous devons donc continuer ce combat, et je souscris pleinement à la demande exprimée par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères de rétablir le comité consultatif franco-japonais relatif à l'enfant au centre d'un conflit parental, qui avait été institué en 2009 et qui avait cessé ses travaux au mois de décembre 2014 à la suite de l'adhésion du Japon à la convention de La Haye. L'instauration de ce comité, tout comme la création d'un poste de magistrat de liaison à l'ambassade de France au Japon, serait un pas important. En effet, pour prendre l'exemple d'un autre pays que je connais bien, je sais combien la mise en place d'un magistrat de liaison français en Allemagne, sur l'initiative d'Élisabeth Guigou, alors garde des sceaux, avait permis une meilleure compréhension du point de vue français en Allemagne. Cette mesure avait considérablement amélioré le traitement de la garde des enfants lors du divorce de couples franco-allemands. Ce dialogue constant entre les deux parties et les mesures récentes prises par le Japon

Pour preuve, le ministre de l'environnement japonais, Shinjiro Koizumi, a annoncé mercredi 15 janvier son intention de prendre un congé de paternité, une décision symbolique qui va à l'encontre des conventions du monde du travail au Japon, mais dont il espère qu'elle donnera l'exemple à tous les pères de l'archipel. Cette évolution lente des mentalités, tout comme notre action, permettra, je l'espère, à l'avenir de mettre un terme à ces drames humains qui brisent les familles. Récemment encore, nous avons pu mesurer, avec deux cas très médiatisés, l'ampleur de ces drames. précédents l'ont évoqué, Louis, âgé de 4 ans, né d'un père japonais et d'une mère française, a quitté Salles-d'Aude le 26 décembre dernier sur décision de justice pour vivre au Japon avec son père. Sa mère a refusé jusqu'au bout de le laisser partir- mes collègues Roland Courteau et Gisèle Jourda connaissent bien ce drame, qui s'est produit dans leur département. Scott McIntyre, un journaliste australien, vient, lui, de passer quarante-cinq jours en détention pour avoir seulement tenté d'apercevoir sa fille et son fils. On peut mesurer les conséquences de ces séparations sur la santé d'un jeune enfant et le traumatisme qu'elles peuvent entraîner à court et à moyen terme. Bien souvent, elles s'accompagnent d'un bannissement total de l'autre culture, de l'autre langue, et et coupent l'enfant de ses racines culturelles. C'est pour tenter de mettre fin à ces drames que le groupe socialiste et républicain votera cette proposition de résolution,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, neuf ans après l'adoption par le Sénat d'une proposition de résolution sur la situation des enfants franco-japonais privés de l'un de leurs parents à la suite d'un divorce ou d'une séparation, force est de constater que que ce dossier demeure toujours très sensible. L'actualité se fait régulièrement l'écho de la détresse de ressortissants français privés de leur enfant consécutive à un enlèvement ou à la non-exécution d'une décision de justice. Des cas de déchirement familial conduisent parfois au pire, certains parents ne trouvant pas d'autre issue que celle du suicide. D'autres risquent la prison en essayant de renouer le lien avec leur enfant, comme ce fut le cas d'un journaliste australien incarcéré après avoir tenté d'apercevoir ses enfants qu'il n'avait pas vus depuis plusieurs mois. Selon l'association Sauvons nos enfants Japon, près d'une centaine d'enfants seraient privés de contact avec leur parent français.

Je salue leurs initiatives pour faire avancer la coopération franco-japonaise sur les droits de ces enfants et de ces parents emportés dans un profond désarroi.

Sur le plan culturel, si la France et le Japon ont en commun le respect des valeurs de liberté et de démocratie, ils n'ont cependant pas la même conception de l'intérêt supérieur de l'enfant. Au Japon, la maison est vue comme entité de la famille et considérée comme un pôle de stabilité sanctuarisé, un point d'ancrage important pour l'enfant, qui doit donc y demeurer coûte que coûte. La justice nipponne s'inscrit dans cette tradition de continuité, héritée de l'ère Meiji qui prévoit, en cas de séparation, que l'un des parents sorte de la famille, donc de la maison. Nos concitoyens concernés par une séparation avec un ressortissant japonais en mesurent concrètement les conséquences. La proposition de résolution le rappelle : le droit nippon de la famille « ne reconnaît ni le partage de l'autorité parentale, ni la garde alternée En France, l'équilibre d'un enfant passe par le lien continu avec ses deux parents, le maintien du contact affectif et relationnel étant considéré comme un facteur du bien-être psychique et moral de l'enfant. Nos juges tentent de le permettre du mieux possible. Ces deux réalités pourraient paraître irréconciliables, d'autant plus que nous sommes tenus de respecter la souveraineté du Japon. Cependant, le Japon a montré des signes d'ouverture. Dans la résolution du 25 janvier 2011, nous appelions Tokyo à adhérer à la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. C'est chose faite depuis 2014. Cette adhésion est censée apporter des garanties en matière de droit de garde et de droit de visite. Comme cela a été rappelé par certains collègues, un espoir se fonde sur la loi relative à l'exécution des décisions en matière civile, adoptée par le Parlement japonais le 10 mai 2019 et qui pourrait améliorer aussi les conditions de la remise de l'enfant au parent détenteur de l'autorité parentale. Malgré ces avancées, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies l'a reconnu, le Japon ne répond pas encore à ses obligations conventionnelles, en particulier en ce qui concerne les déplacements et les non-retours illicites d'enfants, ou encore les cas de déplacement d'enfants à l'intérieur du territoire japonais sans dimension d'extranéité. À cet égard, la présente proposition de résolution évoque à juste titre le défaut d'exécution d'ordonnances de retour en application de la convention de la Haye. Dans l'intérêt de ces enfants, il convient donc d'amplifier les démarches en direction du Japon. La mobilisation du Président de la République sur ce dossier lors de sa visite officielle au Japon, en juin dernier, mérite d'être soulignée.

Nous savons que le Gouvernement oeuvre à la réactivation de cette instance qui a, hélas, cessé de fonctionner en 2014. Enfin, je rappellerai la nécessité de mutualiser les actions diplomatiques avec les pays concernés par la question des enfants binationaux privés de tout lien avec leur parent non japonais. La France n'est pas seule. Le Sénat a adopté, le 18 décembre dernier, une proposition de résolution européenne, dont ma collègue Véronique Guillotin qui va dans ce sens en appelant l'Union européenne à accentuer sa politique de protection des enfants qui se trouvent au centre d'un conflit parental. Mon groupe avait bien entendu soutenu ce texte. Aujourd'hui, animés par le même souci de contribuer à la protection de l'intérêt des enfants binationaux, tous les membres du RDSE approuveront la proposition de résolution qui nous est soumise. Dans un monde de plus en plus cosmopolite où se multiplient les couples binationaux, le droit international et la coopération judiciaire doivent se mettre à la hauteur des enjeux. La parole

Chaque année, des milliers d'enfants sont victimes soit d'un enlèvement international commis par leur parent japonais, soit d'un enlèvement parental à l'intérieur du Japon. Il y a donc urgence à agir, malgré des difficultés certaines. Depuis l'adoption par notre chambre, en 2011, d'une proposition de résolution visant à permettre aux parents français d'enfants franco-japonais de maintenir le lien familial en cas de séparation ou de divorce, il faut reconnaître que le Japon a fait quelques petites avancées. Je pense notamment à l'autorisation de la remise de l'enfant en l'absence du parent ayant perdu l'autorité parentale. Cette loi entrerait en vigueur en avril

plus fortes que la loi. Les lois sont d'ailleurs rarement en faveur des femmes et, dans le cas présent, des mères de famille : ce n'est que mon avis personnel. La seule solution légale, mentionnée très justement

Cet organe permettait de manière effective à des parents, pour des enlèvements perpétrés avant 2014, de retrouver leur enfant et de maintenir un dialogue constant avec les autorités japonaises. Cette mesure s'inscrirait dans la suite de l'installation d'un magistrat de liaison à l'ambassade du Japon en France. Reste donc la voie diplomatique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution européenne déposée par notre collègue Richard Yung a été cosignée par de très nombreux sénateurs de tous bords, comme il l'a souligné lui-même. C'est parce qu'elle fait écho à des situations humaines aussi injustes que dramatiques face auxquelles, quelle que soit notre appartenance politique, nous ne pouvons rester insensibles.

Il n'est en effet plus possible de se taire lorsque les citoyens européens, qu'ils soient Français ou ressortissants d'un autre État membre de l'Union, subissent au Japon des atteintes graves à leurs droits, en particulier quand il est question des droits primordiaux des enfants. Le cas des enfants de parents européen et japonais est un triste exemple : nombre d'entre eux sont maintenus de force au Japon et privés de leur lien avec leur parent européen à la suite d'un enlèvement par leur parent japonais. Certains parents européens se retrouvent en garde à vue, alors qu'ils souhaitaient simplement revoir leur enfant. L'actualité récente a mis en lumière les conditions de détention dans ce pays ! Le Japon ne respecte pas l'accord de partenariat stratégique qu'il a pourtant signé avec l'Union européenne en 2018. Cet accord visait notamment à promouvoir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales. La loi japonaise prévoit, dans le meilleur des cas, un droit de visite de deux heures par mois. Comment peut-on maintenir un lien affectif réel avec son enfant dans ces conditions ? ailleurs, la loi ne prévoit le partage ni de la garde ni de l'autorité parentale, interrompant le lien juridique de l'enfant avec l'un de ses deux parents, et ce au mépris de la convention de La Haye et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, traités que ce pays a pourtant ratifiés. Les ambassadeurs européens ont maintes et maintes fois interpellé les autorités japonaises, le Premier ministre Abe comme le ministre de la justice, sans résultat. La situation est tellement scandaleuse que l'association Sauvons nos enfants Japon a lancé une pétition auprès du Parlement européen, laquelle sera d'ailleurs examinée par les députés européens le 19 février. D'autres initiatives fleurissent de toutes parts pour dénoncer ces situations aussi douloureuses que scandaleuses. Précisons que certains Japonais eux-mêmes ont assigné leur propre gouvernement en justice. En sept ou huit ans, plus de 300 parents français plus de 2 000 parents européens, vivant pour la plupart au Japon, ont fait la douloureuse expérience d'un enlèvement parental dans ce pays. Cela étant, la France a permis à un parent japonais d'exercer ses droits en rapatriant le jeune Louis au Japon contre l'avis de son parent français, alors que l'inverse ne s'est jamais produit lorsque le parent japonais s'y oppose. Je soutiens donc évidemment la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui et dont je suis cosignataire. Elle fait partie des nombreuses initiatives de députés et sénateurs relatives aux enfants franco-japonais victimes d'un enlèvement parental. Notre conseiller consulaire au Japon, M. Thierry Consigny, qui est aussi président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger, attire régulièrement notre attention sur ces drames familiaux. Je m'associe à la détresse des parents et demande qu'un terme soit mis à l'injustice que subissent nos ressortissants français et européens, comme des centaines de milliers de Japonais.

Malheureusement, tragiquement pour nos compatriotes adultes et enfants, la situation n'a pas encore connu d'avancées véritablement significatives. Le sujet est difficile, douloureux et diplomatiquement délicat, puisque nous sommes défavorables à toute proposition renfermant une quelconque injonction vis-à-vis d'un pays tiers. Néanmoins, il nous paraît indispensable que la diplomatie française poursuive ses actions chaque fois que cela est possible, comme cela fut le cas en mai et en octobre dernier. La France a une relation historique privilégiée avec le Japon : nous avons une tradition d'amitié ancienne, précieuse et forte. Cette relation est marquée par une compréhension et un respect mutuels qui doivent nous permettre de dépasser les différences de législation et, surtout, les divergences dans l'application des décisions en matière de droit de la famille. Chacun connaît et mesure la souffrance, le désarroi et le parcours du combattant des pères français empêchés d'exercer leur droit de visite en cas de désaccord avec leur ex-conjointe.

Par ailleurs, il n'existe pas de mesure coercitive en cas de non-respect du droit de visite. De fait, la justice japonaise n'est pas compétente pour intervenir dans ces affaires. Ce n'est possible que si la décision d'exécution est prise par un juge aux affaires familiales japonais, ce qui est très rare, voire inédit, et souvent très onéreux.

que nous ayons en tête les enfants qui se retrouvent privés de leur autre parent, privés de leurs autres racines. Nous ne pouvons pas les abandonner. Ils sont les premières victimes de ces drames familiaux.

sont antérieurs et nécessitent d'autres leviers. C'est aussi le cas pour les déplacements d'enfants à l'intérieur du territoire japonais, sans dimension d'extranéité.

Il importe de créer les conditions d'un dialogue permanent, dans un cadre qui inclurait les spécificités juridiques des deux pays et qui garantirait le droit de l'enfant, conformément à la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Mes chers collègues, je voterai donc en faveur de cette proposition de résolution.

Votre proposition de résolution, monsieur le sénateur, a deux objectifs auxquels le Gouvernement s'associe pleinement. D'une part, il s'agit de s'assurer du respect des droits fondamentaux des enfants franco-japonais au centre d'un conflit parental, dans le respect de la souveraineté du Japon. D'autre part, elle vise à réaffirmer le soutien des parlementaires aux parents français privés de tout contact avec leurs enfants. Je tiens d'emblée à affirmer que cette situation est bien connue du Gouvernement et fait l'objet d'un suivi constant des services de la Chancellerie et du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, que ce soit à Tokyo ou à Paris.

souligné, nous oeuvrons pour que des actions soient menées à l'échelon européen. Je peux d'ores et déjà indiquer que la situation des parents européens privés de contact avec leurs enfants japonais a a été abordée le mois dernier à l'occasion de la réunion du comité mixte chargé de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Japon. Nous avons aussi demandé que cette question soit mise à l'ordre du jour du Conseil de l'Union européenne sur les questions consulaires, afin qu'une stratégie commune soit adoptée. animés que nous sommes de la volonté d'agir, nous serons évidemment très attentifs à l'application dans les mois qui viennent de la nouvelle législation japonaise, qui devrait permettre l'exécution forcée des décisions de justice, en particulier des décisions concernant le retour en France de ces enfants, y compris lorsque le parent japonais s'y oppose. Nous attendrons de la part des autorités japonaises une exécution effective des décisions judiciaires de retour.

C'est pourquoi, de façon plus générale, il nous paraît indispensable de déployer tous les efforts nécessaires pour prévenir et combattre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants, quels que soient les pays concernés. Nous entretenons ainsi des relations et nous organisons des réunions régulières avec les pays avec lesquels nous disposons d'un instrument de coopération, qu'il s'agisse de la convention de La Haye ou de conventions bilatérales. Ces rencontres nous permettent de mener une coopération plus fluide et de régler les difficultés qui peuvent se présenter. Nous avons donc, chaque année, des réunions avec l'ensemble des pays de l'Union européenne pour discuter de questions générales

Enfin, nous organisons des rencontres ou des visioconférences avec l'ensemble des autres pays, soit de façon régulière et institutionnalisée- tel est le cas pour la Russie -, soit en cas de nécessité, par exemple avec Israël, le Brésil, ou le Japon.

Quant à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je sais à quel point vous êtes attachés à promouvoir l'efficacité de la diplomatie parlementaire avec le Japon. Le Gouvernement ne peut que s'en féliciter et encourager les échanges avec les parlementaires japonais sur les évolutions envisageables du droit de la famille japonais qui permettraient de consacrer l'égalité réelle des droits parentaux, ainsi que le maintien effectif des liens familiaux en cas de séparation. Comme plusieurs d'entre vous l'ont indiqué, l'une des principales difficultés tient à l'application du principe de continuité, consacré par le droit et la coutume japonais, selon lequel, lors d'une séparation, un seul des parents est investi de l'autorité parentale. Ce principe conduit malheureusement à exclure l'autre parent de la vie de l'enfant, qu'il soit étranger ou japonais. La société japonaise elle-même s'accommode de plus en plus mal de ce principe, et le gouvernement japonais a récemment lancé une réflexion sur l'introduction possible du partage de l'autorité parentale, voire de la garde alternée. Le ministère de la justice français, comme il a déjà eu l'occasion de l'indiquer lors de la mission conjointe qu'il a menée à Tokyo en mai dernier avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, est tout à fait disposé à partager son expérience avec le ministère de la justice japonais sur ces questions. Je souhaite préciser deux éléments. J'ai noté avec beaucoup d'attention l'invitation faite dans cette proposition de résolution à mieux sensibiliser les magistrats français aux particularismes de ces déplacements internationaux d'enfants vers le Japon. Ces éléments spécifiques pourraient effectivement être intégrés au sein de formations assurées à l'École nationale de la magistrature, sans pour autant vouloir orienter les décisions de nos autorités judiciaires. J'ai par ailleurs demandé à mes services d'expertiser les possibilités d'extension de la zone de compétence du magistrat de liaison de Pékin, spécifiquement pour ce qui concerne l'entrée de civils au Japon. En conclusion, je tiens à réitérer le soutien du Gouvernement à cette proposition de résolution qui vient rappeler ce qui peut paraître une évidence, mais parfois à tort dans les faits

respiratoire aigu sévère) en 2003, l'épidémie du coronavirus qui se profile nous rappelle que les épidémies de maladies infectieuses sont toujours d'actualité ; elles réveillent de vieux fantasmes et conduisent parfois à des réactions totalement irrationnelles. Sans minimiser l'épidémie en cours, je veux simplement rappeler que celle de grippe saisonnière a fait 7 000 morts en France pour l'année 2009, alors qu'on peut se prémunir facilement contre cette maladie trop banalisée. Le changement climatique, en rendant autochtone à la France métropolitaine certaines pathologies jusque-là tropicales, et les grands mouvements de population ne font qu'accroître ces risques, et la seule chose que nous pouvons contrôler est notre capacité de réponse. Encore ne parlerai-je pas des scénarios catastrophes selon lesquels la fonte du permafrost libérerait des virus jusqu'alors congelés, tels que l'anthrax Si, aujourd'hui, une réponse à l'échelon national peut nous permettre, comme nous le voyons, de faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, il m'est apparu pertinent de préciser les dispositions existant en ce sens et de doter notre arsenal d'un niveau complémentaire local. C'est pourquoi j'ai déposé la présente proposition de loi, destinée à encadrer juridiquement de nouvelles méthodes et à équiper au mieux notre pays contre les différentes menaces sanitaires.

sociales s'est montrée soucieuse que les nouvelles mesures de sûreté sanitaire, dont certaines emportent des restrictions de la liberté d'aller et venir pour des motifs d'ordre public, soient assorties de toutes les garanties nécessaires à la protection des droits de nos concitoyens. en ce qui concerne la mesure d'isolement contraint, qui, sans terme explicite, présentait un risque élevé d'inconstitutionnalité. Ensuite, je m'attarderai sur les apports de la commission aux articles 1 à 4, qui renforcent l'efficacité et la pertinence de l'intervention des acteurs publics face aux risques sanitaires émergents que sont les maladies vectorielles, c'est-à-dire transmises par la piqûre d'un moustique porteur d'un agent pathogène. À notre sens, le maire, échelon local de proximité, doit conserver le premier rôle. C'est à lui que doivent incomber la surveillance des zones de sa commune où les gîtes larvaires sont susceptibles de se développer, mais aussi le signalement

la commission a supprimé l'article 3, qui présentait un risque de transfert implicite au maire de la compétence préventive de l'ARS. nous sommes attachés à ce que l'intervention du maire se limite à une obligation de moyens, que constitue le pouvoir de surveillance et de signalement, sans s'étendre à une obligation de résultat, qu'impliquait la fourniture d'états des lieux.

selon que la lutte contre le moustique vise la santé publique ou le confort. La démoustication de certaines zones, historiquement laissée à la discrétion des départements soucieux de développer leur potentiel économique ou touristique, a permis l'émergence d'acteurs spécialisés, d'ailleurs peu connus, dont la compétence doit être préservée. En érigeant la lutte de confort contre les moustiques en compétence obligatoire, l'article 2 entraînait une extension manifeste de compétence à la charge des conseils départementaux

commission que je maintiendrais ma vigilance sur cet enjeu important. Bien que très confiant dans le pragmatisme des professionnels de santé en la matière, je ne suis pas parfaitement convaincu que les dispositions en vigueur assurent une protection satisfaisante de la personne évincée

ont signé un engagement à respecter une quarantaine de quatorze jours, dans un lieu où leur prise en charge administrative et juridique pourrait susciter des inquiétudes. Comment concevoir que cette éviction, à laquelle ces personnes se prêtent pour l'heure sans y être contraintes, ne soit pas assortie de garanties juridiques et financières spécifiques ?

Aujourd'hui comme hier, nos objectifs doivent être à la hauteur des risques. Notre premier objectif est de protéger les populations en nous inscrivant dans une démarche d'amélioration continue du système de santé. de santé. Soyons lucides : la sécurité sanitaire doit répondre à de nouveaux risques, qui se présentent comme autant de défis à relever. Je pense en particulier aux risques infectieux à transmission interhumaine, d'origine alimentaire ou environnementale,

davantage de prévention, de surveillance, de détection, d'évaluation, d'alerte et d'intervention, souvent en urgence. Tel est l'objet de la proposition de loi examinée cet Si le Gouvernement a décidé de la soutenir, c'est qu'elle répond au besoin de renforcer le dispositif de sécurité sanitaire. Les événements que nous connaissons actuellement et ceux que nous avons rencontrés ces derniers mois en confirment toute la pertinence.

Les territoires ultramarins sont régulièrement confrontés à de telles épidémies, mais des foyers ont également été identifiés en métropole ces dernières années. La prévention des maladies transmises par les moustiques, indispensable, nous impose de détruire les gîtes larvaires, notamment en limitant les eaux stagnantes,

pour la sécurité sociale, puisqu'elle s'accompagne nécessairement d'arrêts de travail pris en charge par la solidarité nationale. Rendre la sécurité sanitaire plus efficace, c'est aussi reconnaître qu'elle doit être le fruit d'une action concertée de l'État et des collectivités territoriales. Je pense en particulier au rôle des maires, qui, dans ce domaine comme dans bien d'autres, sont en première ligne face aux angoisses de nos concitoyens. J'en viens aux menaces constituées par des événements naturels ou industriels,

En Auvergne-Rhône-Alpes, l'observatoire régional de santé estimait en 2017 que quelque 650 000 personnes, soit environ 10 % de la population régionale, avaient consommé des soins remboursés en lien avec l'allergie à l'ambroisie, pour un coût global de 40 millions D'autres menaces sont connues, mais elles demandent de redoubler d'efforts pour protéger au mieux nos concitoyens. Songeons aux risques industriels et à la nécessité de compléter les dispositions protégeant les personnes vivant à proximité des centrales nucléaires. la distribution de comprimés d'iode est réalisée grâce à une mobilisation très active des officines de pharmacie, malheureusement, seuls 51 % des habitants concernés vont chercher leurs comprimés.

L'actualité nous rappelle, s'il en était besoin, la nécessité de nous doter de dispositifs adaptés pour éviter la propagation des infections transmissibles. À cet égard, la proposition de loi encadre deux dispositifs préventifs particulièrement nécessaires.

La commission a souhaité s'en tenir aux mesures d'éviction et écarté la possibilité de décréter le maintien à domicile de ces personnes. D'autres pays le font, et nous devons approfondir la réflexion sur le sujet, même si d'évidentes questions se posent en termes de périmètre et de garantie des libertés individuelles. ce qui concerne l'indemnisation des personnes touchées par ces dispositions, nous comprenons l'intention du rapporteur, qui permet de mettre en lumière ces cas particuliers, mais le Gouvernement ne pourra pas être favorable à sa position. Nous en discuterons- c'est tout l'intérêt du débat parlementaire. Des mesures de cette proposition de loi sont attendues par les professionnels de santé, parfois confrontés à des malades qui, ne respectant pas les règles, favorisent la transmission des maladies. Dès lors que les autorités sanitaires et préfectorales sont informées de tels comportements, il convient de leur donner les moyens d'agir dans un cadre précis. À cet égard, le Gouvernement a déposé un petit nombre d'amendements tendant à poursuivre la réflexion entamée par la commission.

en début de semaine qu'une infection par pneumocoque touchait des salariés d'un chantier naval de Marseille, entraînant la mise en place de mesures sanitaires, notamment vaccinales. Citons aussi l'épidémie liée au coronavirus 2019-nCov, identifié en janvier dernier en Chine et, depuis, arrivé en France. Une question demeure : si une réelle épidémie se développait dans notre pays, serions-nous en mesure d'y faire face, et comment ? D'autre part, lors de l'épisode épidémique de bronchiolite hivernale, plusieurs enfants ont dû être transférés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation, faute de lits- reflet du manque de moyens hospitaliers.

À l'évidence, la nette amélioration de la surveillance, de la prévention et de la vaccination a permis de diminuer les risques, voire d'éradiquer certaines maladies infectieuses. Reste que les défis sont multiples pour faire face aux nombreux dangers qui persistent et aux nouveaux qui se profilent.

C'est dire si la veille et l'alerte sont essentielles. Que dire des pathologies potentielles liées aux expositions sanitaires environnementales de notre monde moderne ?

le suivi de cohorte et l'évaluation des expositions. Souvenons-nous de l'amiante et du temps si long écoulé entre les fortes suspicions épidémiologiques et la décision d'éviction de ce cancérogène puissant. Ce cas d'école doit nous rappeler à quel point temps sanitaire et temps des décisions, y compris administratives, doivent mieux converger. Même si nous avons progressé, nous sommes encore loin du compte pour une veille sanitaire efficace débusquant les nouveaux risques. On voit bien que la communauté internationale prend la mesure de l'ampleur de l'alerte sanitaire vis-à-vis des populations. En France, ces sujets nous invitent à revisiter notre organisation, de l'échelle nationale aux échelles régionale, départementale et locale. Cette organisation doit couvrir tous les champs, du signalement à l'alerte, de la prévention à la mise en oeuvre de plans actifs. Tous les éléments de la chaîne de décision méritent d'être évalués, certains d'être améliorés, d'autres repensés, qu'il s'agisse de risques classiques, nouveaux ou émergents plans blancs et rouges, processus de mobilisation de la chaîne administrative et sanitaire, campagnes de vaccination, traitements préventifs, prise en charge médicale, mesures d'isolement et d'éviction, identification et protection contre des facteurs de risques, vectoriels ou non, diffusion de conduites à tenir simples et et compréhensibles pour les citoyens, signalement des cas, recensement dans des registres, réseaux de veille, entre autres. Tous ces sujets sont liés et doivent être traités ensemble, car ils concourent au même objectif.

contacts. Le texte étoffe l'arsenal des mesures mobilisables en cas de risque ou de crise sanitaire. En particulier, il institue des zones de lutte contre les moustiques en vue d'une éradication,

en faisant remonter à l'agence régionale de santé et à Santé publique France les cas de maladies nécessitant une intervention urgente ou une surveillance particulière pour la santé de la population.

Le principe posé est le prononcé de mesures d'éviction : les personnes contacts devront limiter leur présence dans les lieux regroupant du public et relèveront d'un maintien à domicile. L'exception prévue vise à pallier le refus

Reste qu'elle ne nous exonère pas d'une relecture complète de notre système face à l'accélération des événements d'alerte et à l'accroissement de risques nouveaux, différents et aux contours souvent difficiles à définir.

le respect des droits et libertés fondamentales des personnes infectées n'a jamais été aussi prégnante. Il faut dire que l'accroissement des mouvements de population et l'intensification des échanges liée à la mondialisation

à définir la bonne articulation entre l'acteur qui fonde sa compétence sur la proximité de son action, à savoir le maire, et celui qui la fonde sur la spécialité de sa mission, en l'occurrence l'ARS, Si les collectivités territoriales conservent leurs missions d'hygiène et de salubrité, les agences régionales de santé voient leurs missions se renforcer. Ce texte permet donc d'actionner tout un arsenal de mesures, notamment préventives, dont la réactivité et l'adaptabilité sont essentielles pour une lutte efficace contre les maladies à potentiel élevé. les agents habilités auront la possibilité de pénétrer dans les propriétés privées pour mettre en place des actions de lutte en cas de manquement des propriétaires. L'article 4 de la proposition de loi adapte le dispositif de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine pour qu'il ne soit pas exclusivement prohibitif et répressif. la prolifération des végétaux et des insectes nuisibles doit être traitée dans sa globalité, dans le cadre d'une stratégie collective s'affranchissant des limites administratives et géographiques.

Actuellement, deux réglementations concourent à la lutte contre cette espèce : la réglementation sur les dangers sanitaires, mise en oeuvre par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes, mise en place par le ministère de la transition écologique et solidaire. Si la possibilité est désormais donnée aux préfets,

elle réforme notre politique de lutte antivectorielle, sans doute datée, rend possibles de nouvelles mesures d'isolement de personnes contagieuses dans un contexte d'épidémie ou de pandémie, modifie le cadre de la lutte contre les espèces végétales nuisibles, comme l'ambroisie, et tend à assurer une meilleure protection sanitaire des personnes vivant à proximité d'installations nucléaires. Ces objectifs sont louables, compte tenu des risques croissants pour la santé des populations que font peser les grands défis de notre siècle.

Le législateur doit impérativement se saisir de ces problématiques, car notre arsenal juridique y est insuffisamment adapté. La présente proposition de loi répond partiellement

Je ne m'attarderai pas sur les mesures d'isolement de personnes contacts ou infectées prévues aux articles 6 et 7 ; elles font maintenant consensus, dans leur rédaction issue des travaux de la commission. Je serai bref également sur l'article 8, qui prévoit la livraison à domicile de produits de santé nécessaires pour protéger les populations en cas de risque majeur, notamment de comprimés d'iode en cas d'accident nucléaire. Il m'a semblé nécessaire de préciser que cet envoi postal devait être assumé financièrement par l'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage ; au nom de mon groupe, je défendrai un amendement en ce sens. Concernant la lutte antivectorielle, principalement dirigée contre les moustiques, je regrette qu'une telle réforme se fasse au détour d'une proposition de loi, autrement dit sans étude d'impact et sans le travail d'investigation préalable indispensable. Dans ce domaine complexe de l'action publique, un grand nombre d'acteurs Modifier le périmètre de leurs compétences n'est pas anodin. Il ne me semble pas que le législateur soit en mesure de travailler dans de bonnes conditions sans un état des lieux des recherches, notamment entomologiques, médicales et épidémiologiques, sur les dynamiques de propagation des moustiques et des maladies vectorielles associées.

et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles. Cette commission a entamé ses travaux d'investigation en janvier dernier et devrait, dans un délai raisonnable, formuler des recommandations concrètes pour réformer l'intervention publique en la matière. Dans ce contexte, nous craignons que les dispositions prévues aux articles 1 et 2 ne soient prématurées et potentiellement inadaptées. Est-ce une bonne façon de légiférer que de le faire sans avoir tous les éléments en notre possession ? Cela va-t-il devenir une habitude ?

L'article 4 de la proposition de loi ne laisse pas transparaître une grande volonté en la matière. Alors que les associations demandent une territorialisation de la lutte contre l'ambroisie, en associant directement les maires, la logique retenue, qui consiste à calquer le régime juridique applicable à la lutte antivectorielle, me paraît en partie inadaptée et sans doute un peu trop bureaucratique.

ont une grande pratique de la gestion de crise et de l'élaboration de plans techniques, mais trop peu est fait pour que l'échelon local, les acteurs publics comme les populations s'en emparent et se l'approprient. Or, face à un enjeu aussi complexe que la lutte antivectorielle- les gîtes larvaires peuvent se trouver dans n'importe quel recoin urbain où peut stagner de l'eau -, nous ne parviendrons pas à contrôler la situation si nous ne faisons pas confiance à l'échelon local et si nous ne misons pas sur l'implication et la formation des populations. Comme je le disais en préambule, ces enjeux sont non pas les enjeux de demain, mais bien ceux d'aujourd'hui. À cet égard, nous accusons un important retard. Je souhaite que la discussion que nous aurons ce jour permette d'approfondir les différents points cités et que nos amendements puissent contribuer à améliorer encore ce texte, qui est nécessaire. La parole

le travail de Michel Amiel, auteur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Celle-ci vient compléter la loi relative à l'organisation et la transformation du système de santé, que nous avons adoptée l'année dernière. Le texte met l'accent sur les carences dans la gestion de certaines pathologies par les pouvoirs publics et vise à les combler. Il s'agit, d'une part, des maladies vectorielles transmises par les moustiques porteurs d'agents pathogènes, comme la dengue ou la maladie à virus Zika, bien connus de nos territoires, et, d'autre part, des allergies entraînées par la prolifération de certaines espèces végétales nuisibles à la santé de l'homme, telles l'ambroisie. Je vais vais aborder les principales dispositions du texte. L'article 1 réaffirme la répartition des compétences au sein des pouvoirs publics. Tout d'abord, le maire est défini comme étant le meilleur acteur pour repérer ou évaluer le danger d'un événement sanitaire et reste compétent en matière d'hygiène et de salubrité publique. La commission a décidé que son rôle devait être avant tout de signaler, car toutes les communes ne disposent pas de moyens pour lutter efficacement contre un événement sanitaire. En cohérence, l'article 3, qui prévoyait l'obligation pour le maire de faire réaliser un état des lieux en cas de risque, a été supprimé. L'État resterait donc compétent en matière de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, les ARS, qui définissent les mesures de prévention nécessaires, pour le compte du préfet. L'article 4 modifie le régime juridique de la police des espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, afin d'y intégrer un volet préventif.

assouplit le régime de la déclaration obligatoire et supprime la condition de préservation de l'anonymat des données de santé. Il prévoit que les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés puissent signaler à l'ARS les cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale. L'article 6 aborde la question des personnes contacts, présentent un risque élevé de développer une maladie par contact ou exposition, dans des conditions de nature à transmettre cette pathologie et qui doivent limiter leur présence dans les lieux regroupant de nombreuses personnes- personnes- par exemple, des établissements scolaires, des lieux dédiés à l'accueil d'enfants, des lieux de travail ou des lieux de rassemblement. Cette mesure ne pourra excéder un délai de sept jours, renouvelable une fois. Je souscris aux interrogations de M. le rapporteur en ce qui concerne l'indemnisation d'une personne contact évincée. Actuellement, pour pouvoir être indemnisé au titre d'un arrêt de travail, l'employé faisant l'objet d'une mesure d'éviction doit être effectivement atteint de la pathologie justifiant la mesure. Si une personne contact n'est pas contaminée, elle se trouverait, de fait, exclue du champ de l'indemnisation. Or une personne empêchée de se rendre sur son lieu de travail doit pouvoir être indemnisée ! L'article 7 instaure un dispositif spécifique d'isolement contraint pour le cas des personnes atteintes de maladies transmissibles hautement contagieuses qui refuseraient les prescriptions d'isolement, créant ainsi un risque grave pour la santé de la population. Cette mesure d'isolement contraint serait prise par arrêté préfectoral, sur proposition du directeur général de l'ARS, au vu d'un certificat médical circonstancié établi après que la personne aura été mise en mesure de faire valoir ses observations, bien entendu par tout moyen. La commission, soucieuse de garantir l'équilibre entre le maintien de l'ordre public sanitaire et les libertés fondamentales, a notamment décidé de limiter la période d'isolement le temps à un mois renouvelable. Enfin, l'article 8 prévoit que, par dérogation au monopole détenu par les pharmaciens en matière de dispensation au public, la distribution de certains d'entre eux, notamment des comprimés d'iode, pourrait être directement effectuée par livraison à domicile, sous supervision d'un pharmacien.

toutes les communes d'une intercommunalité, dès lors que l'une d'elles entre dans le périmètre du PPI. L'actualité, avec l'épidémie de coronavirus, fait évidemment écho à cette proposition de loi, qui comporte des dispositions

afin d'apporter de nouvelles réponses, plus adaptées, en matière de signalement et de prise en charge des personnes contacts ou infectées. Pour ce faire, ce texte tend déjà à simplifier et à introduire une plus grande fluidité dans les mécanismes de transmission d'informations de santé aux autorités compétentes, avec notamment l'avènement prochain du déploiement intégral du portail signalement-sante.gouv.fr. Ce maillon du signalement de l'information est essentiel pour mettre en place des mesures de prévention de contamination au sein de la population et pour le suivi des personnes contacts ou infectées.

la commission l'a rappelé, l'objectif n'est pas de remédier à un système lacunaire. Il s'agit plutôt de chercher à rendre plus opérationnelle l'action de l'État, alors que les dispositions existantes- je pense en particulier, madame la secrétaire d'État, à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, -semblent présenter l'inconvénient d'avoir défini des habilitations trop larges, donc peu mobilisables. C'est dans le même sens que l'article 6 instaure un réel cadre de prise en charge des personnes contacts. un rapport d'avril 2019, le Haut Conseil de la santé publique rappelle que la personne contact est une personne « ne manifestant pas de signes ou de symptômes de la maladie mais qui a été en contact physique avec un cas (vivant ou mort) ou les liquides biologiques d'un cas pendant la période d'incubation connue de la maladie concernée. » Il rappelle également que, dans le cadre des transmissions interhumaines établies, « les nouveaux cas ont une plus grande probabilité d'apparaître parmi les contacts », d'où l'intérêt de l'article 6.

Actuellement, notre droit ne repose que sur la lutte contre la propagation internationale des maladies. Il convient de prendre en compte les cas autochtones, afin d'étendre le pouvoir de l'ARS agissant pour le compte du préfet. Reste la question de la prise en charge de l'indemnisation des personnes concernées. Je ne doute pas que nous en discuterons dans quelques instants. Enfin, je m'attarderai sur l'article 7, qui prévoit des mesures exceptionnelles pour les cas rares et extrêmes

L'amendement que j'ai défendu en commission et qui a été adopté est inspiré des diverses auditions menées par le rapporteur. Il a permis- là encore, sans s'écarter de l'idée originelle -de préciser plusieurs points : la définition de la maladie pouvant mettre en jeu l'isolement contraint, le rappel que cette mesure doit être motivée et limitée dans son contenu, etc. Cette mesure peut inquiéter par son caractère liberticide, mais elle est équilibrée et permet une plus grande réactivité et une initiative au plus près du terrain pour faire face aux risques liés aux maladies transmissibles hautement contagieuses. Mes chers collègues, l'ensemble de cette proposition de loi doit simplement être envisagé comme une pierre à l'édifice de notre système de santé, dans ses versants de prévention, de lutte antivectorielle et de lutte contre les épidémies.

Cette crise nous rappelle à quel point la prévention et la protection de la population face aux épidémies sont un enjeu de taille pour notre pays. Dans l'exposé des motifs, l'auteur du texte fait le constat de l'insuffisance des moyens d'action nécessaires dont l'État dispose lorsqu'il s'agit de faire face à des maladies infectieuses émergentes de type Ebola sur notre territoire. notre territoire. Dans un premier temps- dans le chapitre I de la proposition de loi -, la responsabilité de l'État pour élaborer et mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles et contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine Ce rappel est essentiel. Nous y souscrivons, raison pour laquelle nous estimons qu'il n'est pas possible de débattre aujourd'hui de ce sujet hors contexte, c'est-à-dire en faisant abstraction des dernières lois relatives à la santé, ont réduit de façon drastique les moyens humains et financiers des hôpitaux, des services d'urgence et de santé en général.

Pourtant, l'hôpital est un service public de premier plan en matière de santé publique. Si le coronavirus atteignait le stade épidémique en France, comment gérerait-on une crise de cette ampleur, alors que les services d'urgence sont à bout de souffle et que les lits sont déjà en nombre très insuffisant ? La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 s'inscrit dans le même schéma : elle est loin d'être à la hauteur des besoins financiers et humains du monde de la santé. de la santé. De même, la loi de finances pour 2020 marque la diminution des crédits alloués à la mission « Santé », sans compter le transfert du financement des opérateurs de santé publique vers l'assurance maladie. La réalité est que l'État se désengage du pilotage financier en matière de prévention et de protection de la santé de la population. Comment analyser autrement le refus opposé par le Gouvernement et sa majorité parlementaire, à l'Assemblée nationale, à un amendement au PLF pour 2020 qui visait à accorder des crédits supplémentaires pour la recherche sur la maladie de Lyme ?

Ces rappels ne sont ni inutiles ni hors sujet. Ils pointent du doigt l'une des interrogations principales soulevées par ce texte l'insuffisance des moyens humains et financiers mis en oeuvre par l'État pour assurer la prévention, la protection et la prise en charge de la population face à une crise sanitaire. Nous savons tous, d'expérience, que, dans ces conditions, la tentation est grande de se défausser de ses responsabilités pour les faire assumer par d'autres : les collectivités territoriales. La proposition de loi, dans sa version première, n'échappait pas à ce travers. Elle porte comme ambition de rationaliser, pour en améliorer l'efficacité, l'intervention des différents acteurs publics. Nous approuvons l'objectif, mais rationaliser ne veut pas dire transférer. Certaines modifications apportées par la commission sont, par conséquent, bienvenues. la suppression de l'article 3, qui transférait une partie des compétences des ARS vers les communes et les maires en matière d'intervention sur les lieux de présence potentielle d'espèces végétales ou animales nuisibles à la santé humaine, sans transfert de crédits ni de moyens correspondants. Nous approuvons également la modification apportée à l'article 2, qui faisait de la lutte contre les moustiques, en tant que nuisance, une nouvelle compétence obligatoire des départements- là encore, sans moyens correspondants. C'est dans le même état d'esprit que nous nous opposons à ce que le coût des interventions des agents sanitaires pour éradiquer des espèces végétales ou animales nuisibles à la santé humaine soit à la charge des occupants des lieux quand leur responsabilité n'est pas en cause. d'une question essentielle et évidente de santé publique. En conclusion, vous comprendrez, mes chers collègues, que, bien que préoccupés par la nécessité d'une meilleure prévention et d'une plus grande protection de la santé de la population, nous ne pouvons que nous interroger sur l'effectivité d'une proposition de loi ne répondant pas à la question cruciale du financement de cette mission par l'État, d'autant qu'une proposition de résolution créant une commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques

la proposition de loi que nous examinons a pour objet de renforcer les capacités de lutte des autorités publiques contre la propagation des espèces nuisibles. Le texte tend à améliorer la résolution de deux problèmes spécifiques de sécurité sanitaire : la propagation des maladies vectorielles, telles que la dengue et le chikungunya, d'une part, et la prolifération d'espèces végétales nocives pour la santé humaine, telles que les ambroisies, d'autre part. L'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement met en lumière l'importance des enjeux en cause dans le cadre de cette proposition de loi. Bien d'autres maladies sont directement concernées par la lutte contre les espèces vectorielles. S'il s'agit d'un problème d'actualité, c'est surtout un enjeu majeur de santé publique. En modifiant les aires de répartition des espèces, le dérèglement climatique nous pousse à nous adapter aux aux nouvelles menaces. Des espèces exotiques migrent ou sont introduites dans des milieux naturels qui n'y sont pas préparés. En parallèle, l'intensification des échanges intercontinentaux accroît la diffusion des maladies. Aussi nous faut-il trouver des réponses opérationnelles aux risques épidémiques et à la prolifération d'espèces exotiques envahissantes. En effet, certaines variétés extérieures déséquilibrent nos écosystèmes au détriment de la biodiversité indigène et nuisent à la santé des populations.

La compétence santé se trouve bien souvent répartie entre plusieurs acteurs. Cette division en fonction des domaines d'expertise de chacun a du sens, mais elle constitue parfois un frein qui ralentit l'action des pouvoirs publics. Nous savons que la salubrité publique relève de la compétence du maire, en concertation avec l'agence régionale de santé. La commission des affaires sociales a souhaité clarifier les champs d'action de ces deux acteurs. Elle a ainsi limité les obligations du maire à un devoir de signalement, et laissé le soin à l'acteur spécialisé qu'est l'agence régionale de santé d'agir à la fois pour prévenir les épidémies et contrôler la bonne exécution des obligations des particuliers. Ces dispositions étaient nécessaires. Elles permettent de délimiter avec précision les domaines de compétence de ces acteurs, dont les interventions gagneront en célérité et en efficacité. La proposition de loi rénove en profondeur l'organisation de la lutte contre les moustiques pour faire face à la recrudescence des cas d'arbovirose propagée par les moustiques et les tiques. Elle clarifie et explicite la compétence du préfet en matière de lutte antivectorielle et consacre l'objectif de lutte contre les moustiques comme compétence obligatoire des conseils départementaux. La commission a souhaité préserver la liberté de décision de ces derniers, en s'opposant au caractère obligatoire de la démoustication initialement prévu par le texte. Dans un contexte budgétaire contraint, nous devons veiller à éviter toute extension de compétence à la charge des collectivités locales qui ne s'accompagnerait pas de compensations financières. Le texte propose également trois nouveaux leviers d'action pour limiter la propagation des maladies vectorielles. Tout d'abord, les procédures de déclaration obligatoire de certaines maladies seront simplifiées, qui permettra une meilleure utilisation de ces dispositifs et en renforcera l'efficacité. Les travaux de la commission ont permis de déterminer que le droit actuel comporte de nombreuses dispositions efficaces dans la lutte contre la propagation de ces maladies. Malheureusement, ces dispositions ne sont actuellement ni utilisées par les professionnels concernés. Ensuite, de nouveaux moyens d'identification des personnes contacts et de prévention de la propagation des maladies seront déployés. Ils sont très utiles pour le suivi des épidémies et nous permettront sans nul doute de renforcer l'efficacité des mesures de prophylaxie. Enfin, en cas d'absence de coopération des personnes contagieuses, une mesure d'isolement thérapeutique contraint par l'autorité sanitaire. Cette disposition a fait l'objet d'un intense travail en commission et son encadrement semble aller vers davantage de respect des droits de chacun, sans toutefois mettre en péril la santé publique. Nous devons rester vigilants quant à la proportionnalité de ces mesures. La liberté d'aller et venir est, en effet, l'une de nos libertés fondamentales les plus précieuses. Sa restriction ne doit intervenir que lorsqu'elle est spécifiquement nécessaire. Nous faisons pleinement confiance au juge judiciaire pour contrôler la légalité d'une telle limitation de la liberté individuelle. Il était important de rendre le droit actuel plus applicable. Ces nouvelles dispositions présentent l'avantage d'être plus opérationnelles et sans doute plus faciles à mobiliser. Les travaux de la commission ont permis de répondre à un certain nombre de difficultés. Le groupe Les Indépendants soutient la finalité recherchée par les auteurs de cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la répétition des épidémies telles que la dengue ou le chikungunya dans les départements d'outre-mer et l'apparition de nouvelles épidémies, comme celle qui est liée font de la sécurité sanitaire un enjeu dont la réalité peut parfois conduire à un véritable traumatisme national. Compte tenu de la présence de vecteurs d'épidémies en métropole, il est essentiel que nous disposions d'un système de lutte antivectorielle efficient. Aujourd'hui, l'actualité législative de notre chambre rejoint l'actualité mondiale. Ce dimanche 2 février 2020, le coronavirus a fait un premier mort hors des frontières chinoises, aux Philippines.

de portée internationale » et de nombreux pays, dont la France, ont annoncé des mesures exceptionnelles. Les personnes à risque, qu'elles soient françaises ou non, ont été isolées sous surveillance militaire à Istres, puis dans un centre de vacances, à Carry-le-Rouet. Or, puisque l'on ne peut pas laisser l'exception devenir la règle, ces mesures exceptionnelles doivent intégrer un cadre législatif qui corresponde aux nouveaux défis qu'impliquent la mondialisation des transports, le réchauffement climatique et la vulnérabilité accrue de nos systèmes immunitaires. Compte tenu de cette dimension internationale des épidémies, les virus ne connaissant pas de frontières, la France doit travailler en concertation avec les autres États membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec les services de l'OMS.

Réunie le mercredi 29 janvier 2020, sous la présidence de M. Alain Milon, la commission des affaires sociales a examiné, sur le rapport de M. Martin Lévrier, la proposition de loi qui nous intéresse aujourd'hui. Celle-ci fait déjà un très large pas dans la bonne direction. D'emblée, le texte réaffirme la répartition des responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales. à l'État d'élaborer et de mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles, sans préjudice des missions d'hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités. C'est, je le crois, sur ce sujet de l'articulation des compétences que doit se porter notre attention la plus vive, en tant qu'élus représentant les territoires, en particulier la ruralité.

Le rôle du maire en matière de lutte antivectorielle doit être limité à un rôle de signalement auprès du directeur de l'ARS, afin de ne pas alourdir excessivement ses missions. La commission a supprimé l'instauration d'une compétence obligatoire de lutte contre les moustiques pour les départements, en raison du coût supplémentaire, important et non compensé, qu'elle impliquait. Elle a également supprimé l'article 3, au motif qu'il présentait un risque de surcharge dans les compétences du maire. Le médecin et l'ARS sont tous deux de bonne volonté. La difficulté réside dans le diagnostic différentiel et le lien numérique entre les deux

à l'ARS- ces signaux faibles constituent en effet le seul outil crédible face aux super-épidémies de demain et à la propagation accrue par la mutabilité des sources et par l'intensification des déplacements. l'article 5 met à la disposition des professionnels de santé des outils informatiques accessibles. Cela dit, parfois, le respect du protocole ne suffit pas. Il faut alors mettre en place des mesures d'éviction, voire de maintien à domicile. concerne l'éviction, il faut généraliser la règle de droit à tous les lieux accueillant des enfants ou de très nombreuses personnes. Pour ce qui est de l'isolement contraint, nous avons décidé de renvoyer à un décret en Conseil d'État ce qui ne relève pas du domaine de la loi. Nous avons garanti la protection des libertés fondamentales par le juge des référés. Nous avons limité dans le temps la période d'isolement contraint à un mois renouvelable. Il faut suivre avec précision le volume d'évolution des cas d'isolement contraint. Sous réserve de cette prudence, je voterai en faveur de ce texte tel qu'amendé par la commission. La parole

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, de prime abord, l'épidémie de coronavirus à laquelle le monde est confronté confirme l'opportunité d'une proposition de loi dont l'objet majeur est de développer un système efficient de prévention des maladies vectorielles-

L'ambroisie constitue une menace directe pour l'homme puisqu'elle est notamment responsable du rhume des foins, de crises d'asthme allergique et de trachéites. Elle constitue également un danger pour les cultures printanières faiblement couvrantes telles que le tournesol.

Compte tenu de leur nature initiale, limitées à des enjeux circonscrits d'hygiène publique et de moralité, les missions de police en matière de salubrité publique ont historiquement fait l'objet d'une attribution générale au maire. Ce dernier, en raison de sa proximité avec le terrain, demeure l'acteur local le plus pertinent

tel qu'il résulte de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, s'entend, à l'égard de l'objet qu'il vise, d'une part, de toute activité de prévention, largement désignée, et, d'autre part, d'une activité de répression plus circonscrite, limitée à la seule « distribution des secours nécessaires La compétence du maire a toutefois été concurrencée, au fur et à mesure de l'expansion et de la diffusion des enjeux de santé publique, par celle d'acteurs spécialisés et déconcentrés de l'État sur les territoires, aujourd'hui les agences régionales de santé. Aussi, l'un des enjeux majeurs de cette proposition de loi consiste à définir la bonne articulation entre l'acteur qui fonde sa compétence sur la proximité de son action, à savoir le maire, et celui qui la fonde sur la spécialité de sa mission, en l'occurrence l'ARS, en matière de lutte antivectorielle.

la compétence de l'agence en matière de lutte antivectorielle. S'il paraît tout à fait normal que le maire se doive de signaler les problèmes, il revient aux ARS et aux préfets d'agir. Je salue ainsi la meilleure coordination entre les compétences attribuées à l'ARS et les pouvoirs des collectivités locales.

Le premier article de cette proposition de loi réaffirme le rôle de l'État dans la politique de prévention des maladies vectorielles. Il est effectivement du ressort de l'État de veiller à la bonne santé de la population. À ce titre, je regrette que le Gouvernement ait décidé de se désengager du pilotage financier de l'Agence nationale de santé publique en faisant adopter dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 une disposition transférant son financement vers l'assurance maladie. Mon groupe avait alors déposé un amendement de suppression de cette disposition qui n'a pas été adopté. Nous n'avons d'ailleurs toujours pas reçu d'explication satisfaisante sur ce point. Toutefois, nous avons une petite idée de la raison ayant présidé à cette décision l'obsession de la diminution des dépenses publiques. La mission « Santé » de la loi de finances pour 2020 a donc vu son budget divisé par deux en prenant également en compte le transfert du financement de l'Agence nationale de sécurité du médicament de santé. Désormais, plus aucun opérateur public assurant la prévention et la protection de la santé de la population n'est soumis au pilotage financier de l'État. De la même manière, l'article 1 renforce les prérogatives des agences régionales de santé, alors même qu'elles subissent également les mesures d'austérité budgétaire ayant conduit à une réduction des effectifs de l'ordre de 338 postes entre 2017 et 2018. Tout cela nous amène à reposer la question de la démocratie sanitaire. Si l'on souhaite que les élus locaux soient pleinement associés et entendus en matière de prévention et de protection de la santé des citoyens sur leur territoire, qu'un grand nombre d'entre eux n'est pas du tout satisfait du modèle soutenu par les ARS pour traiter des questions de santé sur ce même territoire.

Bernard Jomier. Il apparaît nécessaire que le législateur se penche sur l'efficacité de l'organisation actuelle de l'action publique en matière de lutte antivectorielle. Toutefois, cette réflexion doit être précédée d'un certain nombre de travaux. En procédant au moyen d'une proposition de loi qui ne comporte pas d'étude d'impact, nous ne disposons que très partiellement des informations essentielles pour mener sereinement ce travail. Par ailleurs, comme cela a déjà été souligné, l'Assemblée nationale a créé une commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques et des maladies vectorielles. Cette commission d'enquête a entamé ses travaux d'investigation qui portent sur l'évaluation des recherches, notamment entomologiques, médicales et épidémiologiques, sur les dynamiques de propagation des moustiques et des maladies vectorielles associées, sur l'évaluation des politiques de prévention sous leur double aspect- prévention de la propagation des moustiques et prévention des épidémies de maladies vectorielles -et, enfin,

procéder aux opérations nécessaires d'élimination d'espèces nuisibles. Nous connaissons tous l'importance d'une pleine adhésion de la population, surtout au regard de la diversité des gîtes larvaires- une soucoupe pleine d'eau sous une plante est un gîte

Par ailleurs, la référence explicite à l'article L. 1421-2 du code de la santé publique qui prévoit précisément l'intervention de l'autorité judiciaire en cas de refus du propriétaire

cas du malathion, interdit en France depuis 2008 et en Europe depuis 2012, auquel le Gouvernement a accordé un recours dérogatoire en Guyane. Il est nécessaire d'orienter les expérimentations vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement comme celles de la stérilisation de l'insecte, de l'introduction de moustiques au patrimoine génétique modifié, ou encore de l'immunisation des populations de moustiques en les infectant artificiellement par une bactérie les rendant réfractaires au virus de la dengue, par exemple.

en prévoyant que l'exécution des mesures préventives et répressives puisse faire intervenir les communes, les collectivités territoriales mandatées par elles, ainsi que les opérateurs départementaux, fournissent nécessairement l'information préalable à ces acteurs.

défendu. Quel est l'avis de la commission ? Ces trois amendements identiques visent à préciser que les zones de lutte contre les moustiques sont strictement limitées aux nuisances.

allergène dont le rythme de dissémination est élevé, entend améliorer la lutte contre les ambroisies en ajoutant simplement un volet répressif pour les particuliers. la lutte contre la prolifération de ces plantes fait déjà l'objet d'un suivi attentif : arrêté préfectoral sur les mesures à prendre et leur modalité d'application après avis de l'ARS et du conseil départemental de l'environnement ; mise en place de mesures de prévention et de gestion des territoires concernés « clause ambroisie » dans les cahiers des clauses techniques particulières des marchés publics ; nomination d'un référent ambroisie dans les communes touchées.

fois de plus, vous souhaitez vous désengager financièrement de la lutte contre des plantes qui font, comme vous le rappelez si bien, 660 000 victimes et qui entraînent environ 40,6 millions d'euros de frais de santé. La prolifération de l'ambroisie est une question de santé publique. Il revient donc à la puissance publique de s'engager pleinement sur tous les volets, notamment sur celui de la prévention et du coût de la destruction. Nous serions ravis d'en débattre lors du prochain projet de loi de finances. Par ailleurs, cet article prévoit que le coût de l'intervention des agents soit à la charge des occupants des lieux. Nous y sommes opposés. bien d'une question de santé publique, revient-il vraiment aux occupants de payer, quand bien même leur responsabilité n'est pas engagée ni leur négligence avérée ?

sauf dans les cas d'extrême urgence ou de danger, les sapeurs-pompiers n'interviennent plus et la destruction des nids est désormais payante. Aussi, nombre de personnes y renoncent, faute de moyens, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes à court et à long terme en matière de santé publique.

privées. Il faut prendre en compte le fait que le maire, premier échelon de proximité, est susceptible d'avoir à répondre directement auprès de nos concitoyens de l'action de l'État contre les espèces nuisibles. Il est un maillon important de la chaîne d'intervention et doit pour cela être pleinement associé. Il devrait être au coeur d'un système de lutte contre l'ambroisie à la fois souple et territorialisé. Or si la commission a bien fait le choix de renforcer le rôle du maire dans la lutte antivectorielle, ce dernier est absent de la lutte contre l'ambroisie. Je crains même que le dispositif choisi ne retarde l'élimination concrète de la plante en concentrant la décision dans les services de l'État- ARS et préfet de département -, relativement éloignés de la réalité du terrain.

il est essentiel, selon nous, de croiser les approches et de ne pas risquer de mener des actions qui endommageraient les écosystèmes. La lutte contre l'ambroisie est principalement mécanique,

exigences inhérentes à la préservation de la biodiversité en minimisant autant que faire se peut le recours aux biocides. Les alternatives doivent par ailleurs être recherchées, promues et soutenues. Quel est l'avis de la commission

de tout mettre en oeuvre pour éliminer la plante. En cas de refus ou de négligence, elle met en demeure le propriétaire ; puis, dans un troisième temps, l'ARS prescrit que soient exécutés d'office les travaux nécessaires. On peut raisonnablement penser que le délai visé est trop long. C'est en tout cas l'avis des professionnels concernés, car la phase de pollinisation et d'égrainage de l'ambroisie est extrêmement courte. L'élimination de l'ambroisie devrait avoir lieu sous un délai maximal de sept jours, qui est difficilement compatible avec la procédure prévue. Il faudrait donc simplifier

Il s'agit d'attirer votre attention, mes chers collègues, sur la nécessité de rendre toute personne contact évincée, dont je rappelle que la mesure d'éviction la place vis-à-vis de son employeur dans une situation de forte vulnérabilité, éligible au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale. Un décret du 31 janvier dernier a certes prévu des conditions dérogatoires d'octroi des prestations en espèces délivrées par les régimes d'assurance maladie pour les personnes faisant l'objet d'une mesure d'isolement pour avoir été en contact avec une personne atteinte par le coronavirus. Cette mesure n'est toutefois pas satisfaisante ; elle n'est le résultat que d'une habilitation offerte par le législateur, et non d'un droit qui la garantirait directement. Par ailleurs, l'ouverture de ce droit est limitée aux seuls cas de crise ou d'urgence sanitaires, qui ne sauraient, à l'avenir, résumer l'ensemble des hypothèses d'éviction.

n'a d'autre objet que d'intégrer toutes les personnes contacts évincées, quel que soit le contexte général de leur éviction, dans le droit commun de l'indemnisation des arrêts maladie. Quel

actuels liés à l'épidémie de coronavirus. Vous savez que la France a mis en place une stratégie visant à limiter la propagation du virus sur son territoire en assurant la recherche active et la prise en charge précoce des personnes atteintes et de leurs contacts. Une prise en charge est organisée pour les malades, les cas contacts et les personnes ayant séjourné dans une zone où sévit l'épidémie. Ses modalités ont fait l'objet d'une analyse précise du Haut Conseil de la santé publique dans son rapport sur les interventions non pharmaceutiques à mettre en oeuvre pour limiter la propagation des maladies transmissibles lorsqu'il n'existe ni médicament ni vaccin efficace. Le Haut Conseil a retenu trois modalités de prise en charge : l'éviction, le maintien à domicile et l'isolement. nom de considérations pratiques qui tiennent à leur nombre, nous avons choisi de placer à l'isolement dans un même centre d'hébergement nos compatriotes rapatriés. Mais l'objectif prioritaire, rappelé par le Haut Conseil, reste de placer les personnes contacts à l'isolement chez elles ; c'est ce que nous appelons « maintien à domicile ». Ce recours au maintien à domicile est une pratique utilisée par d'autres pays, par exemple le Japon.

comme le port d'un masque, afin de ne pas contaminer leur entourage. L'objet de cet amendement est donc de rétablir, aux côtés de l'éviction qui reste une mesure d'éloignement de premier niveau, la mesure de maintien à domicile qui figurait dans le texte initial de la proposition de loi et dont on voit aujourd'hui toute l'importance. Quel

la crise actuelle à laquelle le nouveau coronavirus nous expose, et en raison des corrections que la commission des affaires sociales a apportées à l'article 6 afin de garantir les droits des personnes évincées, je ne vois pas d'obstacle à ce que la mesure inclue la possibilité de maintien à domicile d'une personne. Avis favorable de la commission.

Gouvernement ? Monsieur le rapporteur, vous soulevez la question de la protection du salarié qui ferait l'objet d'une mesure d'éviction. C'est une question importante puisque, pour des raisons de santé publique, les autorités sanitaires peuvent décider qu'une personne ne se rendra pas sur son lieu de travail pendant plusieurs jours, voire semaines, selon la nature

d'une mesure d'éviction pour motif sanitaire court le risque de se voir reprocher une absence injustifiée par son employeur. La question posée est légitime, et une solution doit être trouvée.

d'État. Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux personnes touchées par une mesure d'isolement contraint en prévoyant que le décret en Conseil d'État qui sera nécessaire pour en préciser l'application devra bien s'attacher à définir les conditions de levée de la mesure.

il convient de circonscrire la dérogation faite au monopole pharmaceutique, en précisant tout d'abord que la liste des produits de santé distribuables par l'exploitant est limitée aux produits de santé « strictement nécessaires à la prise en charge urgente des personnes visées par l'application dudit Par ailleurs, l'exposé des motifs indique qu'il s'agit de prévoir un mode de distribution complémentaire au retrait en officine, ce que le dispositif ne précise nullement. Il est donc proposé d'effectuer Enfin, la mention d'une supervision pharmaceutique est imprécise. Il est proposé de prévoir qu'une convention soit signée entre l'exploitant et un ou plusieurs pharmaciens d'officine, afin de préciser cette articulation.

La supervision de la distribution par un ou plusieurs pharmaciens paraît une garantie suffisante, sans qu'il soit besoin d'y ajouter une convention. Avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis.

une dérogation au monopole détenu par les pharmaciens en matière de dispensation publique des médicaments et de certains produits de santé. Il prévoit également la distribution de certains produits par livraison directe au domicile des personnes. Or la rédaction actuelle ne précise pas l'acteur qui assume la charge financière de cette livraison à domicile. Cet amendement vise à y remédier en prévoyant que cette charge revienne à l'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage concerné.

en cas d'accident nucléaire a été étendu à 20 kilomètres autour des installations. Ces PPI déterminent notamment le périmètre dans lequel des pastilles d'iode sont distribuées gratuitement aux habitants.

à Cattenom, en Moselle. Nos centrales nucléaires sont vieillissantes, et les phénomènes climatiques s'intensifient. Il paraît donc nécessaire d'engager des actions plus poussées en matière de protection sanitaire des populations exposées à ces risques. Si la prise de pastilles d'iode ne permet pas d'éviter l'accident, elle est une solution d'urgence permettant d'empêcher en partie le développement de cancers et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive. Puisqu'il n'est pas question de faire des économies sur la santé de nos concitoyens, et pour répondre à leur inquiétude légitime, cet amendement vise à étendre le périmètre des PPI à l'échelle de l'intercommunalité. L'échelle nationale aurait été préférable, mais nous proposons une solution de compromis : dès lors qu'une commune entre dans le rayon des 20 kilomètres, l'ensemble des communes membres de son intercommunalité intègre également le périmètre du PPI.

L'élargissement de leur périmètre à l'ensemble des communes d'une intercommunalité marquerait un changement radical d'approche en matière de réponse aux risques. Compte tenu de la taille de ces intercommunalités issues des diverses réformes territoriales, de très vastes zones du territoire seraient concernées par ces périmètres. Avis défavorable.